Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.

l'essentiel du temps de parole est réservé aux commissions et, surtout, au Gouvernement, alors qu'il s'agit d'un débat d'initiative parlementaire. J'ajoute que le cadre de ces débats était déjà largement en deçà des exigences démocratiques et pluralistes d'une véritable implication des parlements nationaux dans le débat européen. Or chacun sait que le fossé démocratique qui s'est créé entre les parlements nationaux, les citoyens de chaque pays et les institutions européennes participe de la crise que traverse actuellement l'Union européenne. C'est pourquoi, à l'orée de la campagne des élections européennes et dans un moment où l'Union européenne est confrontée à des problèmes majeurs comme le Brexit, l'accueil des migrants et bien d'autres problèmes qui sont fondamentaux et existentiels pour l'Union européenne et pour les nations qui la composent,

un temps d'explication. Le jeu des questions-réponses est bien sûr très intéressant, mais il conduit à une forme de technicisation de la discussion, si vous me permettez cette formule un peu technocratique. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir donner un souffle au débat

concernant l'organisation de ce débat. Philippe Bonnecarrère l'a très bien expliqué : il ne s'agit pas d'un débat de contrôle ; ce moment s'apparente plutôt à une procédure qui existe au sein de la commission des affaires européennes, au regard

sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler hier, ainsi que sur d'autres dossiers, au conseil Affaires générales, à Luxembourg, en particulier en rencontrant Michel Barnier. La semaine dernière, les négociateurs avaient recherché et cru trouver un équilibre

de maintenir le principe d'une solution de dernier recours, ce que l'on appelle le, qui permette de s'assurer que, si aucune autre solution n'était trouvée, l'Irlande du Nord continuerait à avoir accès au marché unique pour tout ce qui relevait de la mise en oeuvre de l'accord du Vendredi saint et s'alignerait d'un point de vue réglementaire sur l'Union Cette solution aurait été assortie de contrôles aussi facilités que possible entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. En parallèle, l'idée était d'exprimer la disposition des deux parties à négocier une union douanière en bonne et due forme entre l'Union européenne et l'ensemble du Royaume-Uni, limitée dans le temps et qui aurait pris effet après la période de transition. Bien sûr, cette union douanière aurait dû s'accompagner de mesures spécifiques pour s'assurer de conditions de concurrence équitables de part et d'autre de la Manche et de l'assurance d'un accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques. Alors que, vendredi soir, l'accord paraissait atteint, dimanche, les négociateurs britanniques ont fait savoir qu'ils n'avaient pas de mandat politique pour poursuivre dans cette voie. certains expriment aujourd'hui des difficultés à accepter le ; la discussion se poursuit par ailleurs entre ceux qui sont favorables à une union douanière limitée dans le temps et ceux qui la refusent. Mme May sera

comme à l'accoutumée, en présence de Michel Barnier, dont chacun s'accorde à reconnaître qu'il mène un travail exceptionnel. Dans ces circonstances, nous demeurons confiants et déterminés. Ce type de rebondissements n'est pas surprenant dans une négociation aussi importante. Nous restons convaincus qu'un bon accord est encore possible, car c'est l'intérêt bien compris des deux parties. Nous souhaitons donc que les négociations reprennent sur la base du travail technique accompli et que le Conseil européen puisse y revenir rapidement. Le temps presse : conclure un accord dans les prochaines semaines est indispensable, pour que celui-ci puisse être ratifié par le Parlement européen comme par la Chambre des communes.

sur les principes directeurs de la négociation, comme elle a eu à le faire à Salzbourg voilà quelques semaines. Je rappelle ces principes directeurs : dans la relation future, il ne peut y avoir d'accès à la carte au marché unique, de concurrence faussée au détriment des entreprises européennes, d'accès privilégié pour les produits de la mer britanniques si les pêcheurs européens n'ont pas accès aux eaux britanniques, etc. Il faut aussi que Londres accepte toutes les conséquences de l'union douanière si elle prévoit d'y rester et renonce à passer des accords commerciaux en propre. La seconde condition, c'est que nous soyons prêts pour tous les scénarios et pleinement convaincus qu'une absence d'accord demeure préférable à un mauvais accord, comme Mme May nous l'a répété depuis deux ans. Le risque d'une absence d'accord n'étant pas négligeable, j'ai présenté avec Jean-Yves Le Drian, le 10 octobre dernier en conseil des ministres, un projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires en cas d'accord comme en cas d'absence d'accord. Il est de notre responsabilité de nous y préparer. Ce projet de loi d'habilitation demeure général, car nous devrons, dans chaque domaine, nous adapter en fonction de l'évolution de la négociation, négociation, des mesures nationales qui seront prises par les Britanniques et de ce qui sera fait par l'Union européenne pour ce qui relève de sa compétence propre, ainsi que par nos partenaires européens.

mais nous devons faire en sorte qu'un Brexit « sec » pèse le moins possible sur les citoyens de part et d'autre de la Manche et que nous puissions maintenir, autant que possible, la fluidité de nos échanges. Ce projet de loi sera examiné par le Sénat dès le 6 novembre prochain. Au-delà du Brexit, le Conseil européen reviendra sur les questions migratoires. L'enjeu est la pleine mise en oeuvre des conclusions du Conseil européen du mois de juin dernier, dans leurs trois dimensions. Le premier volet est le renforcement de nos relations avec les pays d'origine, mais aussi de transit. développe ses moyens, comme le fonds fiduciaire, et travaille avec les pays d'Afrique du Nord, pour aider ces derniers à mieux gérer les flux migratoires et à mieux poursuivre les trafiquants d'êtres humains. Par ailleurs, la Commission européenne défend un projet nouveau, que nous soutenons, celui d'une alliance Afrique-Europe, pour des investissements et des emplois durables. Le deuxième volet est un meilleur contrôle de nos frontières extérieures, ce qui passe par une forte montée en puissance de FRONTEX, comme le propose la Commission européenne et comme nous sommes en train d'y travailler. Le troisième axe, c'est l'amélioration de nos règles internes, d'abord pour gérer les débarquements. Nous trouvons toujours une solution, comme cela a été le cas tout au long de l'été, et la France prend toujours sa part, mais nous avons collectivement besoin d'un mécanisme européen stable, qui aille au-delà du cas par cas, même si les discussions sont difficiles avec nos partenaires italiens. Nous sommes convaincus qu'une solution durable passe par la mise en place de centres contrôlés en Europe pour assurer une gestion pleinement européenne et solidaire des débarquements depuis le quai. Au-delà, nous devons poursuivre les négociations sur la révision du mécanisme de Dublin et celle de la directive Retour. J'en viens à la sécurité intérieure. Le contexte est particulièrement sensible après l'affaire Skripal et la récente cyberattaque menée contre l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques aux Pays-Bas, dont tout laisse à penser que la Russie et responsable. En matière de lutte contre le terrorisme, nous souhaitons que le Conseil européen donne une nouvelle impulsion politique, afin que les propositions de la Commission européenne soient adoptées, notamment avant la fin de la législature, pour le retrait automatique et immédiat des contenus terroristes en ligne. Nous sommes également favorables à l'attribution au futur parquet européen de compétences antiterroristes. la lutte contre la désinformation devrait être au coeur des échanges du Conseil européen, notamment dans le contexte de la préparation des échéances électorales européennes. Les chefs d'État et de gouvernement se réuniront lors du déjeuner du 18 octobre, en format zone euro dit « élargi ». Il est essentiel de renforcer la mobilisation de nos partenaires, car c'est en période calme, comme nous en traversons une aujourd'hui, qu'il faut mener les réformes qui nous permettront de gérer les crises de demain. Notre objectif est de préparer les décisions que nous espérons voir prises par le sommet de la zone euro au mois de décembre prochain, à dix-neuf, sur la base de l'accord franco-allemand de Meseberg. Cela concerne à la fois l'Union bancaire, la réforme du Mécanisme européen de stabilité et la mise en place d'un filet de sécurité du Fonds de résolution unique, mais aussi la création d'un budget de la zone euro pour la convergence et la stabilisation.

pour que le Conseil européen exprime l'importance d'une très forte mobilisation de l'Union européenne lors de la COP24, à Katowice, au mois de décembre prochain, qui sera un rendez-vous crucial pour garantir l'efficacité de notre action climatique globale.

Si nous voulions en prendre la mesure, l'ordre du jour du Conseil européen auquel vous allez assister, madame la ministre, en est une preuve supplémentaire. Ce Conseil européen devait presque revêtir un caractère historique ; il y a malheureusement peu de chances qu'il en soit ainsi. Je me concentrerai sur deux des sujets que vous avez abordés, madame la ministre, les migrations et le Brexit. La question migratoire, tout d'abord, n'en finit plus de déchirer l'Europe. C'est une onde de choc aux conséquences majeures, qui se fait sentir, scrutin après scrutin, du référendum sur le Brexit aux élections en Italie, en Suède et en Allemagne. L'Union européenne se doit de réagir. C'est un sujet majeur pour les Européens, qui demandent légitimement une meilleure maîtrise de ces flux. Les choses bougent ! Lentement, certes, mais elles bougent : le renforcement la protection des frontières de l'Union européenne est en marche. Des avancées réelles ont été réalisées depuis trois ans, il faut en convenir : renforcement de FRONTEX, durcissement des contrôles aux frontières extérieures, coopération avec les pays tiers ... Le nombre d'arrivées sur le sol européen a ainsi été réduit de 95 % par rapport au pic atteint au mois d'octobre 2015. Pour autant, rien rien n'est réglé. D'une part, sous l'action des trafiquants, les réseaux et les routes se recomposent sans cesse. Les derniers chiffres montrent ainsi une densification des arrivées par la Méditerranée occidentale, mais aussi une reprise des traversées en Méditerranée orientale. Est-ce l'effet d'un relâchement de la surveillance turque ? ? D'autre part, un nombre important de candidats au départ dans les pays sources- particulièrement en Afrique -a l'Europe en ligne de mire. Or, faut-il le rappeler, le continent africain devrait voir sa population passer à 2,4 milliards d'habitants d'ici à 2050. La lucidité et le courage politique nous obligent à dire que le problème de la migration économique et climatique est devant nous, et non derrière La priorité est donc de consolider notre maîtrise des flux. Cela nécessite une action résolue, dans plusieurs directions. Tout d'abord, il faut renforcer la coopération avec les pays de transit du voisinage de l'Europe, ceux de la rive sud de la Méditerranée, pour renforcer leurs frontières. Ce ne sera ni facile ni gratuit, mais il faut poursuivre dans cette voie, qui est efficace : la coopération avec le Maroc est à ce titre exemplaire. C'est en coopérant avec les partenaires du voisinage que l'on trouvera des solutions pour mettre fin à la situation inextricable des migrants qui errent en mer, où, malheureusement, un grand nombre perd la vie. N'allons pas croire que nous pourrons leur imposer des « plateformes de débarquement » dont ils ne veulent pas : c'est une vue de l'esprit, la réponse des pays concernés est bien claire à ce sujet. Dans le même temps, il est nécessaire de poursuivre et d'amplifier notre action en direction des pays sources par l'aide au développement, principalement en matière de maîtrise de leur démographie, mais aussi de la lutte contre les filières d'immigration clandestine. Lorsqu'il y a une volonté, il y a des résultats : l'engagement du Niger, jadis plateforme de tous les trafics, est exemplaire à cet égard. Enfin, un effort significatif doit être fait pour améliorer l'efficacité des politiques d'éloignement des migrants irréguliers. Il y va de la crédibilité de notre politique migratoire. ayons le courage de le dire, nos résultats dans ce domaine ne sont pas encore à la hauteur. Au lieu de progresser, le taux de retour à l'échelle européenne a diminué de 46 % à 36 % en une année. Il est temps de prendre le taureau par les cornes et d'utiliser tous les leviers dont nous disposons pour faire aboutir les opérations de réadmission. Dans ce domaine, nous ne sommes pas totalement dépourvus. Sachons donc être fermes dans notre dialogue -je pense particulièrement aux visas et à l'aide au développement. Des résultats sont possibles pour peu que l'on se mobilise. Madame la ministre, est-ce bien la conviction du Gouvernement ? Est-ce bien sa ligne de direction ? J'en viens maintenant au Brexit, que vous avez évoqué il y a un instant. Je veux saluer tout d'abord l'engagement du Sénat, en particulier du groupe de suivi

Les Européens ont su rester unis au cours des derniers mois. Derrière cette question, vous le savez, mes chers collègues, c'est l'avenir même de l'Union européenne qui est en jeu. Pour la première fois, nous sommes à la veille d'un rétrécissement, d'un amoindrissement de notre projet collectif. Quel non-sens géostratégique !

un impact négatif concret et palpable pour nous tous Européens. Concernant le noeud gordien irlandais, la seule proposition acceptable est aujourd'hui celle du filet de sécurité, ou, que vous venez d'évoquer, la création d'une zone réglementaire et douanière commune entre l'Union et l'Irlande du Nord. Il ne s'agit bien évidemment ni d'annexer ni de réunifier l'Irlande, comme nous l'entendons caricaturer parfois. Nous le savons, ni la réunification ni la réapparition d'une frontière dure ne sont pour l'instant des options possibles. Il nous reste donc à mobiliser toutes nos forces pour convaincre nos amis britanniques qu'une solution est la seule possible. Cette solution doit être flexible, tenir compte de la géographie, de l'histoire et de notre proximité avec le Royaume-Uni. Je veux redire à nos amis irlandais, que nous avons rencontrés avant l'été, que nous serons avec eux dans cette négociation, car nous n'oublions pas qu'ils ont su se montrer solidaires du pack États membres. Le Sénat alerte depuis de longs mois sur les effets désastreux d'un Imagine-t-on une obligation de visa pour les ressortissants de l'Union européenne au Royaume-Uni ou les Britanniques dans l'Union européenne ? Quels droits sociaux, quels accès aux professions après le Brexit ? Les associations de citoyens ne cessent de nous alerter. Nous avions proposé en juillet dernier avec Jean Bizet qu'un protocole séparé soit établi sur cette question, afin qu'elle puisse être réglée quoi qu'il advienne et que les citoyens ne deviennent pas un objet de marchandage. Imagine-t-on, mes chers collègues, l'impact sur les transports aériens, maritimes, ferroviaires et routiers du contrôle sur les marchandises et sur les passagers qu'entraînerait ce ? Les ports français sont en première ligne.

nous serons très attentifs à ce que rien d'essentiel ne soit sacrifié dans le dernier tournant de la négociation et à ce que les mesures qui s'imposent soient prises dans les mois prochains. Madame la ministre, avant votre départ pour ce Conseil européen, nous vous souhaitons bon courage.

Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les présidents, mes chers collègues, si les questions migratoires et de sécurité intérieure occupent la majeure partie des points à l'ordre du jour du Conseil européen, celui-ci est avant tout décisif pour la poursuite des négociations relatives au Brexit. Il sera également l'occasion de réunir un sommet de la zone euro dans une configuration ouverte à l'ensemble des États membres. Ces deux points sont des sujets capitaux pour la commission des finances. Premièrement, alors que l'automne de 2018 avait toujours été présenté comme la date butoir pour parvenir à un accord sur le retrait britannique, ce Conseil européen s'ouvre malheureusement sur l'échec des négociations. La rencontre de dimanche dernier entre le négociateur en chef pour l'Union européenne, Michel Barnier,et le ministre britannique chargé du Brexit, Dominic Raab, n'a pas permis une percée suffisante des négociations. La question persistante de la frontière irlandaise empêche la conclusion d'un accord, alors même que la Première ministre, Theresa May, apparaît contestée au sein de sa propre formation politique. Un accord encore être conclu, mais le calendrier presse en raison des délais de ratification. Or la sécurisation rapide de nos relations futures avec le Royaume-Uni est d'une importance capitale pour notre économie et notre secteur financier. Le Conseil européen de mars dernier a confirmé l'inclusion des services financiers dans le futur accord de libre-échange. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a déjà évoqué par le passé la mobilisation des régimes d'équivalence existants. Comme le rapporteur général de notre commission, Albéric de Montgolfier, l'a rappelé à plusieurs reprises dans le cadre de nos travaux sur la compétitivité des places financières, nous avons estimé qu'il était nécessaire de renforcer l'exigence des régimes d'équivalence. Madame la ministre, pourriez-vous faire le point sur l'avancée des discussions relatives aux services financiers dans le cadre du Brexit ? Plus largement, quels leviers comptez-vous mobiliser à court terme pour assurer la compétitivité de la place financière de Paris ? Plus le blocage des négociations perdure, plus la perspective d'un retrait sans accord devient réaliste. À ce titre, je tiens à souligner l'union sans faille des vingt-sept États membres, qui, depuis le début des négociations, sont parvenus à s'exprimer d'une seule voix pour défendre l'intégrité du marché unique. Les institutions européennes, tout comme le gouvernement français, doivent se préparer à l'éventualité d'un échec des négociations. C'est chose faite pour la France, avec le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce projet de loi d'habilitation contient des dispositions relatives à la continuité de l'utilisation des conventions-cadres en matière de services financiers, indispensables pour la sécurisation de l'exécution de contrats conclus avant la perte du passeport européen par les établissements financiers britanniques. Madame la ministre, le Conseil d'État a émis des réserves sur ce projet de loi et rappelé la nécessité d'indiquer au Parlement le champ de l'habilitation avec précision. Pouvez-vous nous apporter des éléments de réponse à ce sujet ? J'en viens à présent au sommet de la zone euro, qui traitera, une nouvelle fois, de l'approfondissement de l'Union économique et monétaire. Après la publication de la feuille de route franco-allemande, le sommet de la zone euro de juin dernier n'avait malheureusement pas tenu toutes ses promesses. Par conséquent, la gouvernance du Mécanisme européen de stabilité, destiné à servir de filet de sécurité au Fonds de résolution unique, ne sera discutée qu'au Conseil européen de décembre, en raison de la persistance de blocages entre les États membres. Pourtant, le renforcement de l'union économique et monétaire est une priorité pour assurer la stabilité de l'Union européenne. Si le Fonds monétaire international, ou FMI, a relevé en avril dernier les prévisions de croissance de la zone euro pour 2018, il a aussi alerté sur les perspectives de long terme, ce qui nous oblige à « réparer le toit de l'Europe tant qu'il fait beau », selon les termes de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. À ce titre, l'achèvement de l'union bancaire, annoncée depuis de longs mois, doit enfin être concrétisé. La réduction et le partage des risques vont de pair. L'augmentation du ratio de fonds propres des banques et la réduction du taux de prêts non performants au sein de la zone euro témoignent des progrès accomplis pour stabiliser notre système financier. Toutefois, il nous faudra rester vigilants en matière de créances douteuses, notamment dans les bilans des banques italiennes ou chypriotes. De plus, comme l'a indiqué la commission des finances dans une proposition de résolution européenne adoptée il y a bientôt deux ans, la mise en place du système européen de garantie des dépôts ne doit pas se traduire par un par un effort contributif des banques françaises qui pèserait sur leur compétitivité. Voici, madame la ministre, les deux observations que je souhaitais formuler sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire et sur l'union bancaire. Dans quelle mesure, selon vous, le Conseil européen de décembre permettra-t-il de parvenir à un accord et de finaliser rapidement ces réformes ? Enfin, je souhaiterais mentionner les défis à venir pour le budget européen. Alors que le commissaire européen au budget et a appelé les États membres à faire du prochain cadre financier pluriannuel une priorité pour le Conseil européen de décembre, nous pouvons légitimement nous demander pourquoi ce point n'est pas inscrit à l'ordre du jour de demain. La suppression de la contribution britannique au budget de l'Union européenne, ainsi que les désaccords affichés entre les États membres sur les priorités politiques à financer pour la période 2021-2027 font peser des incertitudes sur les orientations budgétaires de l'Union. Comme l'a souligné notre rapporteur spécial Patrice Joly dans ses travaux de contrôle consacrés au cadre financier pluriannuel, l'Union doit se doter de moyens budgétaires à la hauteur de ses ambitions. Il nous faut être vigilants pour que les nouvelles priorités de l'Union européenne ne conduisent pas à remettre en cause la politique agricole Madame la ministre, pourriez-vous nous présenter un état des lieux des négociations relatives au prochain cadre financier pluriannuel ? Alors que l'examen du projet de loi de finances pour 2019 commencera prochainement, pouvez-vous nous indiquer les perspectives d'évolution de la contribution de la France au budget de l'Union européenne d'ici à 2027 ? Par ailleurs, les propositions de la Commission européenne en matière de ressources pour le prochain cadre financier pluriannuel n'ont pas retenu la taxation des entreprises du secteur numérique, alors même que celle-ci pourrait constituer une ressource budgétaire pérenne pour l'Union.

la France a été un moteur dans l'élaboration de cette proposition de la Commission européenne. Êtes-vous optimiste quant à son adoption prochaine ? De quels leviers disposons-nous pour convaincre nos partenaires européens sur ce sujet ? La parole est à M. le président

ce Conseil européen va se réunir autour de trois questions majeures : le Brexit, la crise migratoire et la sécurité intérieure. Ces trois questions portent la marque de l'ampleur des défis que l'Europe doit relever. En premier lieu sera discuté le Brexit. C'est l'occasion pour moi de rendre une nouvelle fois hommage au travail inlassable du négociateur en chef de l'Union, notre compatriote Michel Barnier. Malheureusement, en dépit de progrès réels, la conclusion d'un accord de retrait semble toujours buter sur le problème de l'Irlande. Au travers de son groupe de suivi commun aux commissions des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et des affaires européennes, le Sénat a toujours plaidé pour un retrait ordonné du Royaume-Uni. Il a souhaité qu'une relation étroite puisse être maintenue avec ce grand pays. Le Sénat a aussi lucidement identifié les priorités que l'Union européenne devait impérativement défendre dans la négociation, à savoir le caractère indissociable des quatre libertés de circulation- des biens, des personnes, des capitaux et des services. Celles-ci sont la contrepartie de l'accès au marché intérieur, un marché unique- on ne le répétera jamais assez -, qui est devenu au fil des ans le premier marché économique mondial. Il ne saurait être envisagé de contourner l'indissociabilité des quatre libertés en segmentant par secteur l'accès au marché unique, tant dans l'accord de retrait que dans un accord fixant le cadre des relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Les « difficultés » de l'heure démontrent précisément que nos amis d'outre-Manche n'ont pas tout à fait observé cette indissociabilité. Le groupe de suivi avait aussi clairement indiqué que le Royaume-Uni ne pouvait avoir une position plus favorable en dehors de l'Union que dedans. En juillet dernier, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Le groupe de suivi a pointé le risque de ne pas arriver à conclure dans les temps un accord de sortie ordonnée du Royaume-Uni de l'Union. Faute d'une position de négociation britannique crédible, nous avions fait valoir que l'Union européenne pouvait se retrouver le dos au mur. En particulier, le plan de Chequers s'apparente à un marché unique à la carte, inacceptable pour l'Union. Malheureusement, notre analyse lucide semble se concrétiser.

entre les deux Irlande. La commission spéciale du Sénat examinera avec vigilance et responsabilité le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires

Le dossier migratoire est un autre sujet particulièrement difficile. Nos collègues Jean-Yves Leconte, Olivier Henno et André Reichardt présenteront demain à la commission des affaires européennes un rapport d'information sur l'espace Schengen.

et témoigne malheureusement de la difficulté pour l'Union d'apporter des réponses rapides et coordonnées, alors même que des intérêts essentiels sont en cause. L'Europe est attendue sur sa capacité à protéger ses frontières. Faute d'y parvenir, elle s'expose à de grands risques, qui pourraient se manifester dès les prochaines élections européennes.

Quand les 10 000 gardes-frontières supplémentaires seront-ils opérationnels ? Nous vous posons la question, madame la ministre. Où en est-on concrètement du projet de centres européens contrôlés et des plateformes de débarquement dans des pays tiers ?

de ce sujet, est une exigence humanitaire incontournable et un devoir au regard du droit international, mais l'Union européenne doit aussi agir contre les réseaux de passeurs. Nous devons souligner une nouvelle fois l'urgence de partenariats ambitieux entre les pays d'origine et de transit dans l'esprit du sommet de La Valette. Soyons créatifs au travers de nouveaux mécanismes, à l'image du plan Juncker d'investissements pour l'Europe. En retour, l'Europe doit pouvoir compter sur la coopération active de ces pays en matière de réadmission.

La sécurité intérieure est un autre domaine où la plus-value européenne doit se manifester. Nous l'avons dit au Sénat après les attaques terroristes qui ont frappé la France. Face à des menaces de plus en plus hybrides, la réponse européenne doit d'abord être opérationnelle et intégrer les nouveaux défis, comme la cybersécurité. Il est crucial de renforcer l'échange d'informations et d'assurer l'interopérabilité des systèmes d'information. Peut-on admettre plus longtemps que 85 % des données d'Europol proviennent de cinq pays, dont la France ? Europol doit jouer tout son rôle pour promouvoir la coopération policière européenne. De même, nous appuyons pleinement l'initiative de la Commission européenne tendant à étendre les compétences du parquet européen aux crimes terroristes à dimension transfrontalière.

Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

a affirmé que l'absence d'accord était un scénario plus probable que jamais. La question de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord est bien entendu le point le plus délicat des négociations. dernier, l'Union européenne et le Royaume-Uni s'étaient mis d'accord pour inclure dans l'accord une clause de sauvegarde, sorte de filet de sécurité pour garantir qu'aucune frontière ne soit réintroduite entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Nous sommes favorables à cette option. D'une part, la restauration d'une frontière remettrait en question l'accord de paix du Vendredi saint de 1998, ce qui représente une menace pour la paix en Europe. D'autre part, elle compliquerait la vie des 30 millions d'Irlandais qui traversent la frontière chaque jour. Nous souhaitons un mécanisme de contrôle administratif souple et non intrusif centré sur les marchandises. Ces contrôles pourraient être exercés loin de la frontière, dans les entrepôts ou en mer. Des solutions technologiques existent pour rendre ces contrôles légers, mais efficaces, et il serait souhaitable d'élargir ce type de contrôle souple, pour ne pas léser les entreprises. J'ai cru comprendre que des pays voisins et amis s'y prépareraient.

Mme la ministre.

gouvernements pour négocier avec le Royaume-Uni. Sur la question précise de la frontière irlandaise, nous souhaitons évidemment éviter une frontière dure- nous nous y sommes engagés -et, pour autant, nous protégeons l'intégrité du marché intérieur, puisque la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande est la seule frontière terrestre qui existera entre un Royaume-Uni sorti de l'Union européenne

une progression du réchauffement climatique de 1,5 degré Celsius par rapport à l'aire préindustrielle. Au rythme actuel d'émissions de gaz à effet de serre, ce niveau risque d'être atteint dès 2030.

3 % d'ici à la fin du siècle, engendrant une situation pratiquement invivable pour la moitié de la planète. Pour éviter un tel scénario catastrophe, le GIEC juge désormais absolument impérative une réduction d'au moins

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la sortie prochaine du Royaume-Uni de l'Union européenne impose de s'interroger de nouveau sur le sens de la construction européenne. Les réponses apportées à ce questionnement essentiel déterminent les objectifs de la négociation en cours. Ce débat sur le projet n'est pas sans rapport avec le déclenchement, contre la Hongrie, de la procédure prévue à l'article 7 du traité sur l'Union européenne. En effet, si l'Union est réduite à un marché unique, à une union douanière ou à une association économique, il est alors possible de concevoir une sortie du Royaume-Uni de l'Europe qui préserve l'essentiel des relations commerciales entre les deux entités. De la même façon, si nous acceptons que les valeurs démocratiques constitutives de l'Union soient bafouées par des États membres, alors il faudra se résoudre à accepter que ces pays s'engagent dans d'autres aventures sécessionnistes, renforcés qu'ils seront par la certitude de pouvoir gagner,, eux aussi, un statut qui préserve leurs intérêts économiques essentiels. Jusqu'à présent, l'Union européenne s'est construite sur une logique économique libérale qui a eu pour conséquence de détruire les solidarités sociales et nationales, sans jamais les remplacer par des formes supranationales de cohésion sociale, lesquelles auraient pu lui donner une légitimité politique. Ce double processus de dissociation économique et politique aboutit aujourd'hui à une crise majeure des démocraties européennes qui risque de les mener à l'abîme. Nous ne sauverons pas l'Europe sans le remettre radicalement en cause. Dans l'immédiat, il faut tout mettre en oeuvre pour protéger les accords du Vendredi saint et protéger la paix fragile qui règne dans l'île d'Irlande et ne pas oublier les démocrates de la Hongrie et d'ailleurs, qui ont besoin de l'Europe pour défendre leur État de droit.

Nous ne devons jamais l'oublier. Nous devons également garder en mémoire, lorsque nous parlons de la frontière irlandaise et des accords du Vendredi saint, que la paix a été possible en Irlande du Nord parce que le Royaume-Uni et la République d'Irlande appartenaient à la même Union européenne et parce que l'Union européenne a accompagné la mise en oeuvre de ces accords. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes si attentifs et

Ceux qui ont rédigé le traité de Lisbonne n'imaginaient pas que nous aurions un jour à traiter de cette question à l'intérieur même de l'Union européenne. Pour ma part, je n'imaginais pas, en prenant mes fonctions, que cette question reviendrait aussi souvent au sein du conseil Affaires générales. Hier, nous entendions à nouveau

ailleurs, nous avions un point d'information sur la situation des valeurs fondamentales de l'Union en Hongrie. Il est évident et essentiel que le Conseil se saisisse de ces sujets et qu'il dialogue. L'objectif est non pas de sanctionner

ou tout simplement de sécurité pour les acteurs économiques qui veulent travailler dans ces pays. Tout cela est rappelé de manière régulière. Si nous pointons nous pointons du doigt les violations ou les risques de violations de certains pays, c'est l'attitude de leurs gouvernements que nous déplorons, certainement pas celle des peuples, qui, pour la plupart, restent profondément attachés à l'Union européenne et savent ce qu'ils lui doivent, notamment en matière de politique de cohésion et de solidarité. À cet égard, pardonnez-moi d'être en désaccord avec vous, monsieur le sénateur : l'Union européenne, c'est d'abord un immense mécanisme de solidarité entre les régions les plus riches et les régions plus pauvres,

ils étaient nombreux, deux cent cinquante -et nous avons parlé de l'Europe. Ils vivent dramatiquement ce qui se passe et nous demandent, à nous, politiques, de soutenir un projet dans lequel ils puissent se reconnaître. Ce projet, il le décline très simplement : les droits de l'homme,

Collin. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le Sénat examinera au début du mois de novembre le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Nous aurons sans doute alors l'occasion de discuter, en détail, des conséquences de ce retrait pour notre pays et, bien entendu, pour l'ensemble de l'Union européenne. En attendant, je souhaite évoquer l'une d'entre elles dès aujourd'hui : la perte budgétaire que va représenter le départ du Royaume-Uni,

Dans son relevé de conclusions, le Conseil européen du mois de juin avait pris note de l'ensemble des propositions sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 présenté par la Commission le 2 mai 2018, ainsi que des propositions législatives sectorielles pour les programmes soutenant les politiques européennes. À cet égard, je m'inquiète des moyens alloués à une politique sectorielle en particulier, la politique agricole commune. Mon groupe avait approuvé le 6 juin dernier la proposition de résolution du Sénat en faveur de la préservation d'une PAC forte, conjuguée au maintien de ses moyens budgétaires. Depuis, dans une déclaration commune, dont on peut se féliciter, Berlin et Paris ont demandé « la stabilisation du budget de la PAC L'Allemagne est un allié de poids pour défendre les moyens de la PAC, qui, on le sait, pourraient baisser d'au moins 5 % si l'on s'en tient aux propositions de la Commission.

comme vous, je considère que la politique agricole commune est plus moderne que jamais et qu'elle fait partie de ces politiques ayant une véritable valeur ajoutée européenne. Nous la défendons ardemment

Les négociations commencent à peine. La présidence autrichienne a émis certaines hypothèses, que nous avons immédiatement combattues. J'ai eu l'occasion de le faire hier hier lors du conseil Affaires générales. Au mois de décembre, le Conseil européen se saisira de la question du prochain budget européen. Nous Nous souhaitons évidemment avancer vite mais pas à n'importe quel prix. Nous voulons un bon budget, et pas un budget à tout prix avant les élections européennes. D'autant qu'il nous paraît essentiel que les électeurs puissent s'exprimer sur leurs priorités. Nous devons décliner ces priorités dans un budget, et non l'inverse.

l'autre, une Europe à tendance fédéraliste, qui piétine la souveraineté des États membres pour imposer la pensée unique des pseudo-élites. Plusieurs référendums ont déjà été contournés par les tenants de cette pensée unique, qui n'hésitent pas à bafouer la volonté des électeurs dès qu'elle ne va pas dans leur sens. Aujourd'hui, le Président Macron est à la pointe de la coalition qui essaie de saboter le Brexit en pourrissant la négociation. Là encore, il s'agit de désavouer le suffrage universel en poussant les Britanniques à organiser un nouveau référendum. À la veille des élections européennes, le but est de faire croire à nos concitoyens que l'évolution vers une Europe fédérale est la seule solution possible pour l'avenir. Les responsables ne sont pas de bonne foi lorsqu'ils prétendent négocier des conditions honnêtes de sortie, alors que, dans le même temps, ils exigent la création d'une frontière douanière à l'intérieur du Royaume-Uni pour en disjoindre l'Irlande du Nord. C'est aussi tordu que si, demain, l'Europe demandait à la France de créer une frontière douanière à l'intérieur de notre territoire, par exemple en séparant l'Alsace-Lorraine. Au lieu de chercher à torpiller le Brexit, la France devrait réclamer sa juste part dans la répartition des sièges au sein du Parlement européen. Actuellement, les six députés maltais représentent chacun seulement 69 000 habitants alors que chacun des soixante-quatorze députés français représente 884 000 habitants. Pire encore, en totale violation du traité de Lisbonne, la France a un ratio d'habitants par siège plus défavorable que l'Allemagne. Si ceux qui essaient de torpiller le Brexit parvenaient à leurs fins, cette injustice subsisterait. En effet, lors du Conseil européen du 19 juin 2018, la France a accepté que, en cas d'abandon du Brexit, la répartition actuelle des sièges soit maintenue à notre détriment, et ce en violation du traité de Lisbonne. Madame le ministre, Madame le ministre, pensez-vous qu'il soit acceptable d'organiser les prochaines élections européennes dans ces conditions ? Carrément ! La parole est à Mme la ministre.

et non ceux des Britanniques, comme vous êtes apparemment tenté de le faire ! Heureusement que, pour défendre les intérêts des citoyens et des entreprises européennes,

À l'occasion de ce départ, nous avons pensé à réaffecter les sièges britanniques. Nous avons obtenu, contrairement aux informations qui vous ont été communiquées et qui sont inexactes, de rattraper ce qu'un mandat précédent n'avait pas su défendre, c'est-à-dire le nombre de de députés européens auquel la France a droit. Grâce à cette nouvelle répartition, nous passons à soixante-dix-neuf députés européens français. C'est peut-être l'une des très rares

Mais de quelle sortie parle-t-on ? À J-162 de l'échéance, nous ne savons toujours pas ce que le mot « Brexit » signifie, ou pourrait signifier. À l'évidence, il n'existe pas de consensus au Royaume-Uni en faveur de quelque sortie que ce soit Dans un tel contexte, le mot « Brexit » résonne péniblement pour 5 millions de citoyens européens. Je parle de 3 millions d'Européens qui résident au Royaume-Uni et de 2 millions de Britanniques qui sont installés en Europe. La plupart d'entre eux n'ont pas été appelés à se prononcer sur cette décision. Pourtant, le Brexit les concerne individuellement, intimement. là non pas de tomates, de casseroles ou de véhicules automobiles, mais d'enfants, de femmes et d'hommes. Ils nous interpellent. Les associations qui les représentent font un travail formidable. Je pense à the3million, à ln Limbo ou British in Europe. J'en profite pour saluer l'empathie de notre ambassadeur Jean-Pierre Jouyet à Londres, qui sait les entendre. Le Gouvernement nous a demandé de nous préparer à l'éventualité d'une sortie sans accord. Or les droits des citoyens européens établis au Royaume-Uni, ainsi que ceux des Britanniques vivant en Europe, ont été traités au chapitre 2 du pré-accord de retrait de l'Union européenne, signé en mars dernier. Dans l'hypothèse d'une sortie du Royaume-Uni sans accord, avez-vous prévu, madame la ministre, de préserver cette partie du pré-accord et ainsi de dissocier la question du statut de 5 millions de citoyens européens

y compris en cas d'absence d'accord. J'ai reçu des engagements de la part des Britanniques sur le sort de notre communauté et, plus largement, des communautés européennes au cas où nous ne parviendrions pas à un accord. Vous l'avez très bien dit, la moins mauvaise des solutions se trouve dans l'accord de retrait tel qu'il a été négocié. Nous nous sommes mis d'accord avec les Britanniques sur des mesures protectrices qui permettent à nos concitoyens de vivre, d'étudier, de travailler au Royaume-Uni, dans des conditions comparables à celles qu'ils connaissent aujourd'hui. En cas d'absence d'accord, nous sommes évidemment déterminés à faire en sorte que la période de vie que nos concitoyens passée au Royaume-Uni soit pleinement prise en compte au moment de leur retour en France. Je pense à leurs diplômes, à leurs qualifications professionnelles, à leurs années de cotisations maladie ou retraite. également en sorte que le sort des Britanniques présents sur notre sol soit comparable à celui auquel nous avons pensé dans l'accord de retrait, à une condition, c'est que les mesures prises par les Britanniques, pour nos ressortissants, soient du même niveau. Ma première préoccupation, c'est le sort de nos concitoyens présents au Royaume-Uni. Je tiens à le répéter, la moins mauvaise des solutions figure dans l'accord de retrait. Nous nous efforçons d'obtenir un bon accord.

Cette question est importante pour notre économie locale, en particulier pour les régions littorales comme la Normandie, où les pêcheurs font vivre les territoires tout en respectant les nombreuses réglementations européennes. Attachés à une pêche durable, les pêcheurs s'imposent même des règles de gestion raisonnée, comme pour la coquille Saint-Jacques, afin de préserver la ressource et de garantir des revenus réguliers, règles que les Britanniques ne reconnaissent pas. Vous le savez, le ratissage intense, mais, hélas ! pas illégal, de certaines zones de coquilles, en dehors du cadre défini par la profession, a donné lieu à des affrontements en mer ces dernières semaines. Environ 20 % de la pêche française se pratique dans la zone économique exclusive britannique, sur la base de droits historiques et de la politique commune de la pêche. Ce pourcentage masque des disparités régionales

Aujourd'hui 75 % de la pêche britannique est vendue dans l'Union. Madame la ministre, ma question est simple : quelles initiatives prendrez-vous avec vos partenaires pour préserver les intérêts de la pêche française et européenne, après la période transitoire ou en cas de « ?

négociateurs, ne pourrait être véritablement envisagée qu'à condition que les droits de pêche des pêcheurs européens dans les eaux britanniques soient

n'auraient plus accès aux eaux britanniques. C'est dans cet esprit que nous négocions. Michel Barnier en est parfaitement conscient, je lui en ai reparlé hier, de la même manière que j'en ai reparlé au vice-premier ministre irlandais. L'Irlande, qui est le premier pays

Le Brexit aura donc un fort impact économique et social, y compris dans ce secteur. D'un point de vue politique, cette crise ajouterait encore à la défiance vis-à-vis de l'Europe. En l'état actuel de l'Union européenne, nous ne pouvons nous offrir ce luxe. Tous mes encouragements vous accompagnent aussi, madame.

Les premiers résultats économiques ont été publiés et semblent satisfaisants. On constate ainsi un accroissement significatif des échanges commerciaux et une augmentation des exportations de l'Union européenne vers le Canada de 7 %.

En septembre 2017, la commission Schubert, installée par le Gouvernement, soulignait le manque d'ambition du CETA en matière de protection de l'environnement et surtout l'absence de mesures visant à lutter contre le réchauffement climatique.

du CETA en matière de gaz à effet de serre, l'interconnexion des marchés du carbone et une taxation spécifique du transport maritime. De la même façon, nous attendons, avec toute la société civile, une déclaration interprétative précisant le sens à donner aux dispositions sanitaires et environnementales insuffisamment claires, ainsi que des précisions sur l'application du principe de précaution. L'accord avec le Canada est un accord vivant. Il doit, avant que le Gouvernement nous propose de le ratifier, être amélioré. L'Europe doit exporter ses marchandises, mais aussi ses standards sociaux et environnementaux. Elle doit conclure des accords qui respectent les droits humains et qui préservent la santé, la biodiversité et les équilibres écologiques. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire où en sont les discussions avec l'Union européenne et comment la France entend promouvoir ses standards et faire du respect de l'accord de Paris une condition à la ratification du CETA ? La parole est à Mme la ministre.

l'accord avec le Canada est entré en vigueur de manière provisoire et la Commission a pu faire un premier bilan. Il est très différent de celui que craignaient un certain nombre d'opposants au CETA. au CETA. Cet accord de libre-échange est favorable à nos intérêts, à nos intérêts économiques et commerciaux en général, à nos intérêts agricoles en particulier, contrairement à certaines craintes qui avaient été exprimées. Je note par exemple que les exportations canadiennes de viande bovine à destination de l'Union européenne, loin d'avoir explosé, ont diminué en un an, depuis la mise en oeuvre provisoire du CETA. Cela étant dit, comme vous le relevez à raison,

eurocanadiennes pour la préservation de l'environnement et contre le changement climatique, mais aussi par des mesures bilatérales. Vous l'avez dit,

opposons à la reprise des négociations d'un accord commercial avec les États-Unis, c'est parce que ce pays est sorti de l'accord de Paris. Nous travaillons à titre bilatéral avec le Canada, qui est engagé dans la mise en oeuvre de l'accord de Paris, et nous continuons à négocier avec nos partenaires européens

Pour surmonter les divisions européennes apparues notamment avec l'affaire de l'et ses conséquences humanitaires, les chefs d'État et de gouvernement s'étaient mis d'accord sur deux concepts au mois de juin dernier : celui, d'une part, de plateformes régionales de débarquement, pour le débarquement des personnes secourues dans le cadre d'opérations de recherche et de sauvetage en mer,

vers lesquels seraient transférées les personnes secourues, conformément au droit international. Ces centres devaient permettre de distinguer les migrants en situation irrégulière, qui feraient l'objet d'un retour, des personnes ayant besoin d'une protection internationale. Près de quatre mois plus tard, madame la ministre, où en sont les négociations pour donner un contenu opérationnel à ces plateformes régionales de débarquement ? Où en sont les négociations sur les centres contrôlés ? Plus précisément, la mise en place des plateformes de débarquement requiert la coopération d'États tiers. On a beaucoup parlé de l'Égypte. Pouvez-vous nous donner des précisions sur ce point ? Enfin, la réforme du règlement de Dublin se trouve du règlement de Dublin se trouve aujourd'hui dans l'impasse. La présidence autrichienne souhaiterait éviter de lier solidarité et obligation d'accueil. Quelle est la position française sur ce lien ? Certains pays, on le sait, ne souhaiteraient pas nécessairement avancer sur ce dossier pour des raisons de politique intérieure. Pouvez-vous nous rassurer sur la détermination politique de la France à conclure cette réforme dans les meilleurs délais ? Très bien ! La parole est à Mme la ministre.

introductif sont indissociables les uns des autres et sont le seul moyen d'avoir une politique migratoire européenne équilibrée, efficace et humaine. S'agissant de la question que vous posez sur les plateformes de débarquement, à ce stade, aucun pays du sud de la Méditerranée n'a accepté que de telles plateformes soient installées sur son sol. a formé de grands espoirs s'agissant de l'Égypte et s'est rendue dans ce pays à ce sujet. Il est possible que nous recevions en Europe le Président égyptien pour évoquer plus largement la manière dont les pays du sud de la Méditerranée peuvent nous aider à lutter contre les migrations illégales et comment nous pouvons soutenir leurs efforts, notamment en appuyant leurs gardes-côtes avec du matériel et de la formation. C'est ce qui me paraît le plus prometteur de ce point de vue.

des personnes sauvées en mer. Cette solidarité nous paraît devoir être obligatoire. Les modalités de cette solidarité, elles, peuvent être variables. Mais le principe d'une solidarité obligatoire va de pair avec le maintien d'une responsabilité des pays de premier accueil. Nous avons besoin d'une responsabilité de ces pays de première entrée. Cependant, nous ne pouvons pas les condamner, par leur géographie, à porter seuls l'effort d'accueillir de vrais demandeurs d'asile ayant toute leur place dans l'Union européenne, mais aussi de raccompagner dans leur pays d'origine ceux qui détournent le droit d'asile par souci de migration économique illégale. Ces retours aussi doivent faire l'objet de davantage d'accompagnement européen.

à cette réussite. S'agissant des plateformes de débarquement, madame la ministre, vous l'avez dit, le faible empressement des pays de la rive sud de la Méditerranée à accueillir sur leur sol

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les annexes de l'ordre du jour du Conseil européen comportent des graphiques intéressants sur l'évolution des migrations depuis le début des années 2010

mais une crise de l'accueil, une crise humanitaire, une crise politique interne en Europe. Les maux sont différents, et il faut dire ce qui a été réalisé depuis deux ans sur ce sujet. Aujourd'hui, je voulais vous parler des dix ans de la crise financière, dix ans pendant lesquels les critères de Copenhague, ceux que notre collègue Ouzoulias évoquait au sujet de la démocratie et des droits de l'homme, ont été totalement estompés par une version dure des critères de Maastricht, c'est-à-dire une exigence d'austérité budgétaire qui s'est imposée à l'ensemble de l'Europe. La crise financière de 2008, pour cette raison, a fragilisé voire cassé l'image d'une Europe

depuis le début de ce débat ; c'est cela qui pèse sur l'image de l'Europe aujourd'hui ! Pourtant, l'union économique et monétaire n'est pas parachevée ; l'union bancaire est bancale. Ainsi, on a harmonisé les règles de protection des dépôts en Europe,

avec quelle gouvernance ? une gouvernance intergouvernementale non démocratique, comme les propositions du sommet de Meseberg, ... Cher collègue ! ... ou avec le Parlement européen, pour superviser ce nouveau budget et son exécution ? La parole

mais la mutualisation des dépôts reste un sujet difficile. Naturellement, le budget de la zone euro est un sujet essentiel, sur lequel nous sommes parfaitement engagés, convaincus. La déclaration de Meseberg était un pas en avant très significatif puisque, conformément au contrat de coalition, le gouvernement allemand a appuyé l'idée d'une capacité budgétaire de la zone euro à la fois pour l'investissement et pour la stabilisation. Nous sommes donc allés aussi loin que nous pouvions le faire. Demain, à l'heure du déjeuner, nous allons évoquer les progrès de la réforme de la zone euro, essayer de convaincre nos partenaires qu'il faut le faire maintenant, sans attendre qu'une situation internationale, qui n'est pas aussi stable que certains le pensent et peut être troublée, nous y force. S'agissant de la gouvernance, je partage votre point de vue et nous souhaitons un Parlement de la zone euro ou,, une formation du Parlement européen dédiée

lient d'une manière ou d'une autre leur propre monnaie à l'euro. Mais nous devons faire plus pour permettre à notre monnaie unique de jouer pleinement son rôle sur la scène internationale disait, voilà quelques semaines, Jean-Claude Juncker. Paradoxalement, en Europe, 80 % des factures d'importation d'énergie sont réglées en dollars américains, alors que seulement 2 % de ces importations proviennent des États-Unis, et certains pays européens vont jusqu'à acheter des avions européens en dollars. Pourtant, depuis sa mise en circulation le 1 janvier 2002, l'euro s'est affirmé comme une devise internationalement reconnue, notamment en matière de monnaie de réserve, juste derrière le dollar qui conserve, nous le savons, une position dominante dans le bilan des réserves de change des banques centrales, mais aussi en tant que monnaie de règlement des transactions commerciales, où il fait désormais presque jeu égal avec le dollar. Toutefois, cela a déjà été évoqué, l'euro n'est pas encore reconnu comme un instrument d'investissement,

Madame la ministre, à l'heure où l'extraterritorialité du droit américain, fondée notamment sur l'usage du dollar, menace de sanctions des entreprises européennes et, plus largement, la souveraineté diplomatique des pays membres de l'Union européenne et de la zone euro, je reviendrai, comme un certain nombre de mes collègues, sur la nécessité de renforcer cette union économique et monétaire de la zone euro et d'achever l'union bancaire et l'union des marchés de capitaux. merci. l'euro doit être, comme le dollar, une monnaie de référence, vous l'avez dit, et la zone euro est une puissance économique équivalente à celle des États-Unis ou de la Chine. L'euro est d'ores et déjà la deuxième monnaie la plus échangée dans le monde. Ainsi, 36 % des paiements internationaux étaient réalisés en euros en 2017, mais nous avons à l'évidence une importante marge de progression. L'exemple que vous donniez tout à l'heure était, de ce point de vue, éclairant, et ces 36 % ne reflètent pas le poids de la première économie mondiale. Vous l'avez dit, dans son discours sur l'état de l'Union européenne, le 12 septembre dernier, le Président Juncker a indiqué vouloir développer davantage le rôle international de l'euro,

sans doute sous la forme d'une communication. Nous serons évidemment très attentifs aux propositions qu'elle pourra formuler à cet égard. Vous avez raison de le souligner, il y a un lien évident avec les sanctions américaines, puisque les autorités américaines considèrent qu'elles peuvent sanctionner toute entreprise, même étrangère, qui utilise le dollar. Je me réjouis que la résolution européenne du Sénat sur les moyens de contrer l'effet extraterritorial des sanctions américaines ait mis cette dimension en avant.

Mme Fabienne Keller. Madame la ministre, je reviendrai sur le sujet du Brexit. Plus les négociations avancent, plus, vous l'avez rappelé, madame la ministre, la perspective d'un « » se précise, et je salue votre anticipation à travers le projet de loi d'habilitation à prendre des ordonnances que vous avez déposé. Comme vous le savez parfaitement, si l'on ne s'y prépare pas, l'absence d'accord pourrait avoir des conséquences dramatiques pour l'Irlande du Nord.

la concurrence loyale et nos intérêts, notamment en matière de pêche, ou bien nous en revenons au filet de sécurité qui avait été agréé au mois de décembre et qui est, comme me le confiait hier le vice-premier ministre

ni le rétablissement d'une frontière ni la réunification de l'île d'Irlande ne sont des hypothèses sur lesquelles nous travaillons. Il faut donc trouver une autre solution.

Mme Laurence Harribey. Madame la ministre, ma question lie l'une des priorités inscrites au prochain Conseil européen, la question migratoire, et un volet qui sera sans doute prioritaire dans le Conseil européen du mois de décembre, le budget. le budget. Pourriez-vous faire le point sur le chantier relatif au programme européen destiné à soutenir les collectivités locales accueillant des réfugiés, un fonds envisagé en 2015 et proposé en avril 2018 devant le Conseil européen par le Président de la République Cette proposition soutenue par un certain nombre de parlementaires européens, notamment français, allemands et portugais, permettrait de prendre en compte la dimension territoriale

européen. Au sein de la politique de cohésion de l'Union européenne, qui consiste à lutter contre les inégalités, à accompagner ceux qui en ont le plus besoin, une aide aux collectivités territoriales qui accueillent des migrants et des réfugiés nous paraît s'imposer comme un instrument permettant de financer du logement, de la formation, de l'accompagnement pour les personnes nouvellement arrivées sur le territoire européen. Au lieu d'être une politique de sanctions contre ceux qui n'accueillent pas, c'est une politique d'encouragement pour ceux qui le font. Nous savons d'ailleurs que ces propositions ont recueilli un écho jusque dans certaines communes de certains pays dont les gouvernements se disent hostiles à l'accueil des réfugiés politiques. Nous portons donc cette proposition au sein du prochain budget européen. Les négociations sont en cours. La parole est est à Mme Laurence Harribey, pour la réplique. Je voudrais simplement insister sur l'importance de ne pas lâcher sur cet aspect de la question. Vous avez souligné l'importance d'une gestion européenne et solidaire de la question migratoire : c'est vrai sur le plan intergouvernemental, mais c'est indispensable aussi sur le plan local, pour tenter de freiner l'exploitation de cette question par les populismes en tous genres.

dans le monde, le nombre d'enfants migrants voyageant seuls a été multiplié par cinq depuis 2010. Selon l'UNICEF, au moins 300 000 enfants non accompagnés ont été enregistrés dans quatre-vingts pays en 2015. L'Europe n'est pas à l'abri de ce phénomène, puisque l'on estime qu'en 2016 un demandeur d'asile sur trois avait moins de dix-huit ans et 63 000 demandes d'asile d'enfants isolés ont été enregistrées dans l'Union européenne. Comme vous le savez, ces mineurs qui prennent la route vers l'Europe sont particulièrement vulnérables. Être parvenus jusque sur le territoire européen ne met pas fin à leurs problèmes, car, au sein même des États membres, les normes et les pratiques nationales ne suffisent pas à garantir leurs droits, voire contreviennent parfois aux impératifs de protection. Les procédures de détermination d'âge, les conditions d'accueil, les formalités varient d'un État à un autre. L'Italie, par exemple, enregistre un nombre d'arrivées qui n'a cessé de croître. Mon département, les Hautes-Alpes, enregistre depuis 2015 un nombre exponentiel de mineurs non accompagnés provenant majoritairement du continent africain, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. en 2015 à 2 028 dossiers en 2018, alors que l'année n'est pas terminée ! Cette situation est sans précédent pour le conseil départemental des Hautes-Alpes. L'aide sociale à l'enfance a dû faire face à l'hébergement d'urgence de ces jeunes gens qui se déclarent tous « mineurs » lorsqu'ils arrivent et, par conséquent, à des évaluations en très grand nombre. À ce jour, cette situation très disparate entre les États membres fait la part belle au trafic humain et des filières se sont organisées afin d'acheminer ces jeunes jusqu'aux frontières nationales

politique d'aide publique au développement qui permette d'offrir de véritables perspectives dans les pays d'origine. Naturellement, les routes qui sont empruntées par ces mineurs

dans sa politique de développement, avec une part de 0,38 % de son revenu national brut, qui doit monter progressivement à 0,55 % d'ici à la fin du quinquennat. C'est là, à travers des réponses très concrètes liées à à l'auto-entrepreneuriat, à l'investissement dans des microentreprises, des petites entreprises que nous arriverons à donner un espoir et un avenir à cette jeunesse pour lui éviter ces traversées de la mort.

La parole est à M. Christophe Priou. Monsieur le secrétaire d'État, parmi les trois chantiers européens pour organiser la maîtrise du phénomène migratoire, la sécurité des frontières extérieures, l'harmonisation de la politique des États membres et la réduction des incitations à la migration irrégulière, il me semble utile de revenir sur la question de la sécurisation des frontières européennes. Le mandat confié à l'Agence européenne FRONTEX pour contrôler les frontières de l'Union européenne n'est certainement pas à la hauteur des enjeux. Là comme dans bien d'autres domaines, hélas, l'inertie européenne risque de nous coûter cher à l'arrivée et de nourrir les populismes, l'Union européenne n'étant pas en mesure d'assurer la fouille, la saisie, le déroutement ou la destruction des navires utilisés en haute mer pour le trafic des migrants dans les eaux territoriales libyennes, ni de lutter contre les passeurs et de neutraliser leur chaîne logistique pour empêcher le départ des bateaux de migrants. La lutte à la source est largement en deçà des besoins : seuls 110 passeurs ont été arrêtés depuis 2015. Malgré un renforcement du budget de FRONTEX, près de 340 millions d'euros en 2018 contre 143 millions en 2015, son efficacité reste à démontrer, avec 1 300 agents sans équipement propre propre et sans pouvoir réel. La situation devrait évoluer d'ici à 2020, il en a été question vendredi dernier à Luxembourg. Mais, une fois de plus, l'Union n'anticipe pas les crises ; elle les subit. Plusieurs pays restent réticents à l'idée de faire des gardes-frontières européens une force en mesure de déployer ses effectifs aux frontières de l'Union. Compte tenu des moyens limités pour contrôler les frontières extérieures, je ne suis pas certain que le souhait de la Commission européenne appelant vendredi dernier à mettre fin à la prolongation des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen soit de nature à rassurer tous les membres de l'Union européenne et leurs peuples.

dans la solidarité, mais aussi dans la responsabilité, qui est d'allouer des moyens humains, financiers, budgétaires, là où le besoin s'en fait cruellement ressentir.

Plusieurs pays de l'Union européenne craignent pour leur souveraineté puisque l'agence FRONTEX a vocation à assumer des responsabilités dévolues aux États. On constate une nouvelle fois, hélas, que l'Europe ne parle pas d'une seule et même voix.

L'âge des enfants non accompagnés est une question décisive pour leur assurer une protection et leur offrir des garanties dans le contexte de la migration. Il s'agit en effet d'un processus très complexe ayant pour but de définir le régime juridique applicable à un individu qui peut être lourd de conséquences pour celui-ci. Or, parmi les obstacles juridiques opposés à la prise en charge immédiate des enfants isolés, figure en première ligne la tendance constante des administrations des États membres à contester leur minorité, soit parce qu'ils n'ont pas de papier certifiant leur état civil, soit parce que l'authenticité de ces papiers est remise en cause. En effet, les méthodes appliquées pour définir l'âge de l'enfant diffèrent d'un État membre à l'autre, et les procédures d'évaluation ne sont pas toujours fiables. Il n'existe actuellement aucune procédure d'évaluation, qu'elle soit médicale ou autre, permettant de déterminer sans marge d'erreur l'âge exact d'une personne. Ces disparités peuvent se traduire par une série d'incidences négatives pour les enfants, telles que faire l'objet d'une erreur d'identification en tant qu'adulte ou être placé en rétention avant et pendant le processus de détermination de l'âge. Les enfants qui ne sont pas reconnus comme tels risquent d'être laissés en marge du dispositif. Outre le risque qu'ils n'accordent pas à un enfant la gamme des droits qui sont les siens, certains processus de détermination de l'âge peuvent même, dans leur conception et leur mise en oeuvre, traumatiser ces enfants déjà bien vulnérables. À cela s'ajoute la gravité des résultats de l'évaluation pour les personnes qui en font l'objet et les répercussions potentiellement potentiellement néfastes du processus sur leur santé physique et mentale, ce qui souligne la nécessité d'élaborer des lignes directrices, dans le cadre relatif aux droits de l'homme, applicables à la détermination de l'âge. Je me dois de rappeler que les conséquences d'une mauvaise estimation ... Il faut conclure, ma

la Commission estime justement que la différence et la variété des régimes existant dans les différents pays européens ne permettraient pas de dégager de lignes

La France, au travers, notamment, de son action en matière d'aide publique au développement, parce que tout est lié, accompagne un certain nombre de gouvernements et d'États

mené sur ce sujet pourrait permettre d'apporter une réponse dans le temps, structurelle, au sujet que vous posez. De ce point de vue, je peux vous assurer de la détermination intacte du Gouvernement, comme l'indique le nombre de projets qui se multiplient dans le cadre de cette aide au développement.

du Conseil de l'Europe, qui défend les droits de l'homme et la démocratie, et il m'apparaît comme absolument indispensable et nécessaire de trouver une coordination entre les États et les diverses autorités, pour respecter les droits de ces enfants. Pour conclure

que nous nous orientons. Dont acte. Chacun prendra ses responsabilités, il faudra être pragmatique et intelligent. Mais ce n'est absolument pas ce que nous aurions souhaité.

travaille sur cette question. Le concept de développement durable doit être au coeur de la solution à ce problème, à terme. Autrement dit,

un étiquetage des produits de pêche britannique, nous y viendrons et je suis persuadé que le consommateur européen saura faire la différence. Très bien ! Monsieur le secrétaire

les Pays-Bas, la Belgique, sont véritablement, au travers de leur administration, aux côtés de leurs entreprises nationales. Cela veut dire précisément

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en procédure accélérée, du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

M. François Bonhomme. Les mineurs d'aujourd'hui ne sont plus ceux de 1945 ; c'est une évidence. Le cadre légal de la justice des mineurs doit donc être adapté pour en tenir compte. les auteurs de cet amendement souhaitent restreindre l'excuse pénale de minorité applicable aux jeunes âgés de seize à dix-huit ans. En effet, les mineurs de plus de seize ans représentent près de la moitié des mineurs impliqués dans des affaires pénales. La nature des actes qu'ils peuvent commettre justifie donc qu'ils fassent l'objet de sanctions proportionnées et dissuasives.

beaucoup plus fourni, si je puis me permettre cette expression. Il ne s'agit pas de nier que la problématique soulevée par les auteurs de cet amendement est une problématique réelle, dont il faut aujourd'hui tenir compte, j'allais presque dire malheureusement. Quel

a érigé au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs- c'est une décision de 2002.

est à M. François Bonhomme. Afin de permettre au juge d'adapter la peine sans recourir à l'emprisonnement ou à des sanctions éducatives de moindre portée, cet amendement prévoit que la peine consistant en l'exécution de travaux d'intérêt général, actuellement limitée aux mineurs de plus de seize ans, peut être prononcée à partir de l'âge de treize ans. Entre treize ans et seize ans, les parents devront donner leur accord préalable.

monsieur le rapporteur, madame la ministre,

Cet amendement vise à favoriser la réinsertion des jeunes ayant commis des faits relevant de la petite délinquance, par le biais d'un encadrement militaire volontaire. Il est d'ailleurs inspiré par les services des armées prenant en charge les jeunes déscolarisés.

Il s'agit d'un système incitatif, dès lors que ces jeunes volontaires bénéficieront d'une réduction du délai d'effacement de leur casier judiciaire, s'alignant sur la durée maximale du service, à savoir un an ou huit mois, au lieu de trois ou cinq ans. Un tel dispositif est de nature à responsabiliser les jeunes délinquants en quête de réhabilitation du fait de la nature volontaire d'une inscription à ces types de service militaire. Par ailleurs, la nature de cet encadrement leur permet de renouer directement avec le respect de l'ordre et de la discipline, ainsi qu'avec le sens du dévouement envers le bien public. Enfin, le but de ce service militaire étant de favoriser l'insertion professionnelle, cet encadrement a vocation à permettre à ces jeunes de se réinsérer durablement dans la société. En Île-de-France, ce sont près de 72 % des jeunes engagés au sein de ce service qui sont insérés professionnellement. À travers cet amendement, j'entends ainsi consacrer un droit à l'oubli pour des jeunes ne demandant qu'à se reconstruire une vie digne et honorable, par le biais de l'effort et du travail. Quel

Il existe actuellement deux modalités principales de réhabilitation : soit une réhabilitation de plein droit, qui a lieu après l'exécution de la peine principale ; soit une réhabilitation après une décision judiciaire. Les auteurs de l'amendement envisagent de créer un nouveau cas de réhabilitation, évidemment au-delà de l'absence de nouvelles condamnations dans certains délais. dans certains délais. En cas de condamnation unique à une peine de prison qui n'excède pas un an ou à une peine d'une autre nature que de l'emprisonnement, dès lors que l'intéressé n'est pas en état de récidive légale, ils proposent que la réhabilitation puisse être acquise si, après l'exécution de la peine, la personne concernée réalise un service militaire volontaire d'une durée de douze mois ou un service militaire adapté d'une durée de huit mois.

un contrôle du juge sur la sortie de la délinquance d'une personne condamnée, il me semble indispensable que s'écoule une certaine durée entre la condamnation d'une personne

en touchant aux règles de réhabilitation légale, qui permettent l'effacement d'une condamnation du B2 du casier judiciaire. Les condamnations prononcées contre les mineurs ne figurent pas au B2, seulement accessible aux administrations ou à certains organismes privés. Globalement, je suis donc défavorable à cet amendement, pour des raisons à la

Depuis mars 2012 et les attentats de Toulouse perpétrés par Mohammed Merah, la France a subi une quinzaine d'attentats, avec un bilan effroyable : plus de 240 morts, victimes de la folie et de la haine islamistes. Dans la plupart des cas, les terroristes kamikazes y ont aussi laissé leur vie, et rares sont ceux qui ont pu être interpellés afin d'être jugés. C'est cependant le cas de Salah Abdeslam, seul rescapé du commando du 13 novembre 2015. Si son procès est attendu, de nombreux Français ont appris avec stupéfaction que cet individu allait bénéficier de l'aide juridictionnelle pour payer sa défense. Même s'il s'agit là d'un cas heureusement rare, nous ne pouvons que nous interroger sur le bien-fondé de l'exercice de ce droit pour les auteurs d'actes terroristes. En effet, les actes terroristes ne sont pas des crimes et des délits comme les autres. À travers leurs victimes, les terroristes s'attaquent aussi et surtout à une société, à une civilisation et à une vision de l'humanité. Nous sommes tous attachés à la notion d'État de droit. Mais, de même que la liberté d'expression n'autorise aucunement à dire ou à écrire n'importe quoi, le principe de l'aide juridictionnelle ne saurait être dévoyé. saurait être dévoyé. En donnant corps, en 1972, à l'aide juridictionnelle, qui permet à tous les citoyens, quel que soit leur niveau social, d'avoir accès à une défense juridique, les législateurs avaient-ils imaginé que ce droit servirait un jour les intérêts d'un terroriste ? Il est permis d'en douter, surtout lorsque l'insolvabilité supposée de l'accusé est totalement contradictoire avec les moyens dont il a bénéficié pour échafauder ses projets meurtriers. Aussi, par souci de défense des intérêts de la Nation et de la cohésion sociale, je vous propose, avec la quarantaine de cosignataires de cet amendement, de retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux auteurs d'actes terroristes ainsi qu'à leurs complices.

sur un plan strictement juridique, qu'un tel amendement pourrait être considéré comme contraire à nos principes et valeurs constitutionnels, contraire au principe d'égalité, contraire au principe du droit à un recours juridictionnel effectif, contraire au principe de l'exercice des droits de la défense,

Je ne suis pas persuadé que répondre à la barbarie par un État de droit qui commence par nier la nécessité de se défendre soit ce qu'attendent nos concitoyens. Une société doit avant tout reposer sur un pacte social, ce que l'on appelle le « contrat républicain ». Ce qu'attendent avant tout nos concitoyens, c'est

il y ait le procureur, les magistrats de la cour d'assises spéciale, composée uniquement de juges professionnels, et une défense, qui n'est pas là forcément pour soutenir l'action du terroriste, mais pour garantir l'équité du procès.

On ne peut pas soupçonner Jean-Pierre Grand d'être le complice de ceux qui veulent abattre la démocratie ou de ceux qui voudraient être trop généreux ou trop indulgents avec les terroristes. Mais, de grâce, mes chers collègues, nous sommes

d'interventions de nos collègues, de notre rapporteur et de Mme la garde des sceaux, qui m'ont paru très convaincantes et pertinentes. Je voudrais dire aux auteurs de cet amendement que tout accusé est présumé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. La question ne devrait donc même pas se poser : nous ne pouvons pas punir quelqu'un en lui refusant un avocat pris en charge par l'aide juridictionnelle avant de savoir s'il est coupable. Et nous ne pouvons pas savoir s'il est coupable s'il n'a pas été défendu au cours d'un procès. Supposons qu'une cour d'assises se réunisse. L'accusé, poursuivi pour complicité d'attentat terroriste, clame son innocence. Au cours du procès, coup de théâtre il a été pris pour un autre ... La cour d'assises est convaincue de son innocence et le relaxe.

lui. Simplement, dans un État de droit, on ne peut pas mettre en prison, parfois à perpétuité, quelqu'un qui n'a pas été défendu. Et si cette personne n'a pas les moyens d'assurer sa défense, l'aide juridictionnelle doit évidemment être appliquée. Ce n'est pas faire preuve de complaisance à l'égard des terroristes que de rappeler cette règle fondamentale de notre État de droit. Monsieur le président

mettre en place un système de frais de justice pour assurer le financement de l'aide juridictionnelle. Je rappelle que la loi du 29 juillet 2011 avait instauré une contribution pour l'aide juridique forfaitaire de 35 euros. À l'époque, il s'agissait de financer l'obligation pour l'État d'indemniser des avocats commis d'office

l'article 52 vise à rétablir la contribution pour l'aide juridique, supprimée par la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Elle serait désormais modulée, de 20 à 50 euros, en fonction du type d'instance engagée. À l'instar du dispositif supprimé, ladite contribution n'aurait pas à être acquittée pour certaines matières contentieuses, auxquelles cet article ajoute les procédures engagées par les salariés devant les conseils de prud'hommes. Les personnes éligibles à l'aide juridictionnelle ne seraient pas non plus redevables de la contribution. N'y a-t-il pas là une contradiction, voire quelque chose de choquant ? Non seulement cette disposition constitue une entrave financière non négligeable à la charge du justiciable, mais ce financement complémentaire de l'aide juridictionnelle tend à faire peser sur les seuls justiciables les moins fortunés le fonctionnement des institutions judiciaires. Ce n'est pas notre vision de la justice.

Comme l'ont rappelé nos collègues, la contribution pour l'aide juridique avait été supprimée en 2013 par le projet de loi de finances pour 2014, au motif que, depuis sa création, en 2011, elle avait découragé des justiciables à aller en justice. Comme l'estimait la Chancellerie en 2013, « les contentieux de faible montant, comme les injonctions de payer, ont connu une diminution des saisines du juge de l'ordre de 13 % entre le premier semestre de l'année 2011 et le premier semestre de l'année 2012. Cette baisse, contemporaine de l'introduction du timbre à 35 euros, laisserait présumer que celui-ci constitue un obstacle à l'accès au juge, à tout le moins dans les petits litiges dont le gain escompté est faible. » Il nous semble que ce constat, valable en 2013, doit continuer continuer d'être regardé comme tel en 2018 : une réintroduction de la contribution pour l'aide juridique aurait des effets en premier lieu sur les petits litiges, ce qui s'oppose à la recherche d'une justice de proximité.

Elle serait désormais modulée de 20 euros à 50 euros, en fonction du type d'instance engagée. Ce droit de timbre existe actuellement en cause d'appel, son montant étant de 225 euros. Le rétablissement de cette contribution, qui rapportait chaque année à peu près 50 millions d'euros aux caisses de l'État, a le mérite d'apporter une réponse simple, pérenne, efficace aux difficultés permanentes de financement de l'aide juridictionnelle, dont les dépenses sont en augmentation continue, continue, pour un coût limité pour le justiciable, grâce à la modulation prévue par le dispositif que nous avons intégré dans le texte. Comme lors de sa mise en place en 2011, cette contribution n'aurait pas à être acquittée pour certains contentieux, auxquels cet article, d'ailleurs, ajoute les procédures engagées par les salariés devant le conseil des prud'hommes. Par ailleurs, comme par le passé, les personnes éligibles à l'aide juridictionnelle ne seraient pas non plus redevables de cette contribution. Quel est l'avis du Gouvernement

a introduit un nouveau titre qui vise à accroître la maîtrise des dépenses d'aide juridictionnelle. C'est évidemment un objectif que partage pleinement le Gouvernement, mais, pour autant, nous n'avions pas nous n'avions pas décidé d'inclure dans cette loi de programmation et de réforme de la justice des dispositions sur l'aide juridictionnelle. Je redis ici ce que j'ai eu l'occasion de préciser devant la commission qui m'a entendue il y a évidemment une difficulté, que je qualifierai de pérenne, autour de la notion d'aide juridictionnelle, qui tient à sa construction. Nous avons donc décidé de demander un rapport à l'Inspection générale de la justice et à l'Inspection générale des finances. Ce rapport, qui vient de nous être rendu, évoque

le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et la Bâtonnière de Paris, de prendre le temps du dialogue et de la construction d'un dispositif pérenne autour de ce projet. C'est la raison pour laquelle, volontairement, nous n'avons pas mis de dispositions à ce sujet dans le projet de loi que je vous présente. je vous présente. Cependant, je vous indique que nous avons budgété pour l'année 2019 des provisions suffisantes pour, d'une part, évidemment, maintenir le paiement de l'aide juridictionnelle dans les conditions dans lesquelles elle fonctionne aujourd'hui, et, d'autre part, prévoir également une augmentation liée à l'accroissement de la représentation obligatoire qui est prévu dans le projet que je vous propose. Nous avons donc sécurisé les financements

je me pose plusieurs questions. D'une part, je m'interroge sur la précision de cet article au regard du principe d'égalité devant les charges publiques, dans la mesure où aucun critère n'est défini pour déterminer le montant de cette contribution au sein de cette fourchette de 20 à 50 euros. Il y a donc un doute sur une question juridique. D'autre part,

conçu comme une manière de responsabiliser les justiciables dans leur présence au sein du service public de la justice en les sensibilisant sur le coût réel de la justice et sur les saisines abusives. Toutefois, le paiement des frais de justice

de vote. En 2014, Jacques Mézard et moi-même avions rendu un rapport sur l'aide juridictionnelle, dans lequel nous avions pris acte de la suppression du droit de timbre,

Il me semble qu'il y a là une contradiction majeure. Chacun sait bien que la justice n'est pas gratuite, en réalité, et que le droit de timbre est simplement une contribution solidaire pour l'accès de tous à la justice. Il faut autoriser cette contribution, qui permettra de régler bien des problèmes

l'amendement n° 42. Cet article, qui a été introduit par les rapporteurs du texte, s'inspirant d'une mesure adoptée par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi sur le redressement de la justice, prévoit que toute demande d'aide juridictionnelle est précédée de la consultation d'un avocat, lequel vérifie que l'action envisagée n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. Selon nous, cette mesure porte atteinte au principe d'accessibilité de la justice, en ajoutant un obstacle supplémentaire au parcours du justiciable qui souhaite saisir la justice, mais qui n'en a pas les moyens. Par ailleurs, confier aux avocats, qui sont des acteurs privés, une mission relevant de l'autorité de l'administration, dans le seul objectif de réaliser des économies, n'est pas admissible. Rappelons que « la justice est la sanction des injustices établies », pour reprendre les mots d'Anatole France, qui devraient nous inspirer.

juridiques. Dans le rapport que Jacques Mézard et moi-même avions rendu, nous avions prévu le contrôle de la recevabilité au fond de l'affaire par le bureau d'aide juridictionnelle dans sa composition pluripartite.

Je vais évidemment vous présenter une série d'amendements de suppression pour les raisons que j'ai indiquées précédemment, à savoir que je ne souhaite pas introduire de dispositions sur l'aide juridictionnelle. Soit je détaille à chaque fois les raisons pour lesquelles je souhaite la suppression, soit on considère que ma position est liée à la problématique générale,

l'amendement n° 300 rectifié. Comme cela vient d'être dit et comme cela a été évoqué lors de l'examen de la proposition de loi pour le redressement de la justice, la réforme proposée pour le contrôle de l'attribution de l'aide juridictionnelle rendant obligatoire la consultation préalable d'un avocat pose de nombreuses questions de principe et de mise en oeuvre. tend à faire porter sur les avocats la charge d'un contrôle aujourd'hui effectué par l'administration, un contrôle qui devrait, au contraire, être renforcé, comme vous le proposez par ailleurs, messieurs les rapporteurs. D'autres l'ont déjà souligné, il s'agit également d'un obstacle supplémentaire entre le justiciable et le juge. C'est pour ces raisons C'est pour ces raisons que nous y sommes opposés.

des actions pour lesquelles le justiciable est défendeur ou, en matière pénale, des demandes relevant de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle en raison de leur caractère urgent. Il s'agit de rendre effectives les dispositions prévues à l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 1991 relative à l'aide juridique, qui n'a jamais été appliqué en pratique. Cet article prévoit que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. Bien sûr, la mise en place de cette mesure supposera une organisation spécifique des barreaux, ainsi que divers ajustements pratiques qui devront être réglés par le pouvoir réglementaire. Ce dispositif, s'il fonctionne correctement, devrait améliorer grandement le contrôle de l'attribution de l'aide juridictionnelle. Cette attribution obéit aujourd'hui à une logique de guichet, disons les choses telles qu'elles sont 90 % des demandes formulées en première instance donnent lieu à une admission, alors que ce taux est de 23 ,5 % en cassation, où l'aide juridictionnelle est refusée aux demandeurs si aucun moyen de cassation sérieux n'est relevé. Un grand nombre de rapports ont été rendus ces dernières années sur ce sujet-là,

par les rapporteurs de vouloir assurer un meilleur contrôle de l'attribution de l'aide juridictionnelle, cet article sous-entend que certains justiciables feraient la demande de l'aide juridictionnelle alors que leurs ressources seraient suffisantes pour se payer les services d'un avocat par leurs propres moyens. donc proposé de récupérer les informations nécessaires pour juger du bien-fondé des demandes en sollicitant les organismes de sécurité sociale et les organismes assurant la gestion des prestations sociales. Cette logique de suspicion à l'égard des plus vulnérables n'est pas acceptable, d'autant moins lorsque l'on connaît les difficultés que rencontrent les personnes les plus précaires pour accéder aux informations concernant leurs droits en matière d'aide juridictionnelle.

afin de permettre aux bureaux d'aide juridictionnelle d'avoir accès aux données mises à disposition par la CNAF et qui sont nécessaires à l'instruction d'une demande d'aide juridictionnelle, notamment le service « Mon compte partenaire ». Pour toutes ces raisons, il me semble que la modification de la loi proposée par la commission n'est pas nécessaire.

Mme la garde des sceaux. L'article 52 vise à confier l'ensemble de la procédure de recouvrement de l'aide juridictionnelle au Trésor public. L'État peut recouvrer les sommes versées aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle auprès de la partie adverse, quand celle-ci perd son procès. Dans ce cas, on utilise la procédure de recouvrement de recettes non fiscales. Les états de recouvrement sont adressés au cours d'appel, lesquelles transmettent ensuite les titres de recettes au service du Trésor public. L'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de la justice, dans le rapport dont je fais état depuis maintenant quelques amendements,

selon elles, ne serait pas pertinent. La direction générale des finances publiques a fait évoluer son dispositif de recouvrement des recettes non fiscales pour plus d'efficacité. Elle a confié le recouvrement comptable de l'ordonnateur qui émet le titre de perception. Il me semble que cela devrait améliorer le taux de recouvrement. Nous allons également, comme je l'ai déjà dit, développer un nouveau système d'information pour gérer l'aide juridictionnelle, ce qui devrait faciliter l'identification des sommes à recouvrer. Je demande donc la suppression de l'article

juridictionnelle à la suite d'une décision de retrait de l'aide ou auprès de la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès, dès lors que celle-ci n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en confiant ce recouvrement au Trésor public, dont on connaît la capacité « à faire ». En pratique, le retrait de l'aide juridictionnelle n'est que très rarement ordonné, puisqu'il représente environ 0,1 % du nombre annuel d'admissions. Et quand il l'est, les sommes ne sont recouvrées que dans 3 % ou 4 % des cas.

En effet, des personnes qui auraient individuellement les moyens de se pourvoir en justice, notamment à l'encontre de l'administration dans le cadre de recours contre un permis de construire, utilisent une association

De tels abus, à mon sens, ne sont pas acceptables et constituent un véritable détournement de l'esprit de la loi. Dès lors, il est proposé de limiter ces abus en conditionnant l'accès des associations à l'aide juridictionnelle

des associations soient prises en compte pour apprécier si elles sont éligibles à l'aide juridictionnelle. Cette proposition nous pose deux difficultés. D'une part, son application est limitée aux actions devant les juridictions administratives, alors que les dispositions de l'article 2 de la loi de 1991 concernent les règles relatives à l'attribution de l'aide juridictionnelle devant toutes les juridictions.

au nom et dans l'intérêt de l'association, et non pas au nom de tel ou tel membre en particulier. Il est donc difficile, pour ne pas dire compliqué, de faire supporter les frais du procès aux membres de l'association qui auraient du patrimoine. Dans ces conditions, je sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable.

ces actions ont tendance à proliférer. Vous me dites qu'il n'est pas possible de procéder ainsi, mais il ne faut pas s'étonner ensuite si des associations voient le jour à cette seule fin.

Sur le fond, je soutiens sa démarche. Néanmoins, je suis sensible à l'argument du rapporteur par rapport aux deux ordres de juridiction. Limiter cette

représentation obligatoire par avocat, et donc un coût supplémentaire pour l'aide juridictionnelle. Cependant, le texte adopté par la commission et par le Sénat n'ira pas tout à fait dans le même sens. Par ailleurs, madame la garde des sceaux, vous nous avez annoncé une réforme tirant les conséquences de réflexions en cours,

créativité et ingéniosité des agents des juridictions qui, face aux contraintes budgétaires, parviennent néanmoins à faire de nécessité vertu ! Ces initiatives doivent être valorisées et méritent d'être examinées. Une initiative particulière a retenu notre attention, qui va dans le sens d'une justice de proximité, la délocalisation partielle et ponctuelle des services de greffe dans des territoires du ressort éloignés des juridictions et moins bien desservis.

de la commission ? La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. En premier lieu, si le tribunal de première instance comporte plusieurs sites, en remplacement des anciens tribunaux d'instance, il y aura nécessairement des fonctionnaires de greffe à demeure dans ces sites.

qui devrait distraire un certain nombre de moyens humains dont la nécessité est aujourd'hui établie dans les tribunaux existants. En cinquième et dernier lieu, le ministère de la justice peut décider de localiser des greffes détachés, donc permanents, dans certains sites,

mais il a existé des greffes détachés seuls et on pourrait en recréer demain. Toutefois, la formule n'a pas rencontré, il faut le reconnaître, un grand succès compte tenu de l'isolement des fonctionnaires concernés. Il faut aussi mentionner la présence d'un greffier dans un grand nombre de maisons de justice et du droit, qui devraient, à terme, rejoindre les SAUJ, les services

de l'article, entendait déjà mettre en place la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance avec la création de « chambres détachées », qui ont pour vocation de remplacer les tribunaux d'instance vidés de leur substance, le texte de la commission va encore plus loin en réintroduisant les « tribunaux de première instance », les TPI. Aussi, alors que le Gouvernement n'excluait pas de conserver plusieurs tribunaux de grande instance sur un même département, il s'agit ici de consacrer le principe du tribunal unique par département, sous couvert de la complexité qu'engendrerait la spécialisation à l'échelle départementale. Nous sommes opposés à la création de ces tribunaux. qu'elle ne répond en aucun cas au souci de proximité du justiciable avec les lieux de justice, d'autant que chacun connaît la disparité de nos départements. Il suffit, pour

Le souci de proximité sera d'autant moins respecté que les chambres détachées semblent n'avoir été pensées que dans l'optique de supprimer ensuite, sans rencontrer grande opposition, les sites de tribunaux d'instance.

claires, précises, préétablies et stables, afin d'éviter que le juge ne soit choisi en fonction des affaires. Or « le risque est important que les juges dont les décisions juridictionnelles auraient déplu plus prompts que d'autres à la contestation des décisions de leur hiérarchie héritent des situations les plus inconfortables », dénonce le Syndicat de la magistrature. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. La seule logique pécuniaire et gestionnaire guide ces mesures, au détriment de la justice de proximité et de l'égal accès au droit pour tous les les justiciables de notre pays. Cela vient d'être dit, je ne vais pas gloser beaucoup plus, il est beaucoup plus facile de fermer une chambre détachée qu'une juridiction. La ruralité est quand même aujourd'hui en grande difficulté. Elle se heurte à des problèmes de transports, à des fermetures de commerces, d'écoles, de services publics. Le service public de la justice doit continuer à être accessible.

le projet d'évolution de l'organisation territoriale que je porte pour la justice. Comme j'ai eu l'occasion de l'affirmer à plusieurs reprises, je souhaite une justice plus simple, plus lisible et plus efficace pour les citoyens, une justice qui s'adapte aux évolutions de notre société tout en restant

La commission des lois du Sénat a compris cette ambition, d'une part, en votant, comme je le proposais, le regroupement administratif des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance et, d'autre part, en renonçant

La commission des lois souhaite introduire une nouvelle dénomination en créant un tribunal de première instance. Je ne partage pas ce choix parce que, selon moi, dans l'esprit de nos concitoyens, le tribunal de première instance renvoie à l'idée de tribunal départemental, que j'évoquais précédemment et que je ne souhaite pas créer. Il me semble nécessaire, sur ce point, de lever une certaine ambiguïté.

demain, le justiciable n'aura plus qu'une entrée unique, par une requête unique, devant le tribunal, quel qu'il soit, qu'il s'agisse du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, d'un tribunal d'instance isolé ou bien d'un tribunal d'instance regroupé au sein du tribunal de grande instance, comme cela se passe d'ailleurs aujourd'hui dans beaucoup de villes moyennes. Ces

garanti par décret. Ce socle de compétences comprendra l'ensemble des compétences dévolues aux anciens tribunaux d'instance, notamment

la consommation, des baux d'habitation et des tutelles, de tout ce qui forge le contentieux du quotidien. La création de ce juge des contentieux de la protection viendra

La prise en compte de ces fragilités mérite en effet une affectation dans les tribunaux de proximité, comme au siège des tribunaux de grande instance. J'observe au passage que votre commission des lois m'a rejointe pour partie en créant un juge des tutelles et un juge des contentieux de proximité. Je propose, pour ma part, un juge unique prenant en charge l'ensemble de ces dossiers. Votre commission des lois m'a rejointe, mais pour partie seulement,

Eh bien, il me semble que nous devons, dans certaines hypothèses, rendre cette spécialisation envisageable pour nos magistrats. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé

mon projet a évolué pour tenir compte des craintes exprimées par les avocats et les territoires. J'ai donc décidé que ces compétences spécialisées ne pourraient porter que sur des compétences techniques, d'une part, et de faible volumétrie,

Votre commission m'a rejointe sur un certain nombre de points. Je pense notamment à mon idée d'ouvrir la possibilité de confier à l'un des procureurs, dans les départements qui en comptent plusieurs, un rôle de coordination des politiques publiques judiciaires sous le contrôle du procureur général. Il s'agit là aussi

cet amendement, qui est contraire à notre position, je fais un point général. La commission a approuvé le principe de la fusion entre le tribunal de grande instance et les tribunaux d'instance de son ressort, sans remise en cause de la carte judiciaire, ni création d'un tribunal unique par département, tout en conservant les sites des anciens tribunaux d'instance, en dehors du siège de cette nouvelle juridiction unifiée sous forme de chambre détachée. Le socle des compétences des chambres détachées serait fixé nationalement, par décret. Des compétences supplémentaires

Le Gouvernement avait envisagé, dans un premier temps, de garder la dénomination de tribunal d'instance pour les chambres détachées, ce qui nous paraissait une source de confusion. Le Gouvernement propose à présent la dénomination de « tribunal de proximité Or, outre que cette dénomination donne l'impression de recréer les juridictions de proximité supprimées depuis plusieurs années, on ne peut pas donner à ces sites judiciaires le nom de « tribunal », car ils n'en sont plus. De plus, comment comprendre la coexistence d'un tribunal de grande instance sans tribunal d'instance et d'un tribunal de proximité qui n'est pas vraiment un tribunal ? Ce choix sémantique serait sans doute pour certains justiciables une source de confusion. Il est faux de dire que le tribunal de grande instance est bien identifié aujourd'hui, sinon nous ne ferions pas la réforme Sur cette question de dénomination, le Gouvernement a fait état d'un problème constitutionnel. Il ne paraît pas que l'argument soit recevable, il relève plutôt du nominalisme juridique. On ne pourrait pas réformer les tribunaux de grande instance ou seulement modifier leur dénomination au motif que l'article 65 de la Constitution évoque la nomination des présidents des tribunaux de grande instance par le Conseil supérieur de la magistrature. Dans ce cas, comment le Conseil supérieur de la magistrature peut-il statuer, aujourd'hui, sur la nomination des présidents des tribunaux de première instance dans les collectivités d'outre-mer du Pacifique, alors qu'ils ne sont pas formellement cités dans la Constitution ? De plus, pour répondre aux incertitudes sur la carte judiciaire, la commission a voulu mettre en place un dispositif encadrant toute modification du siège ou du ressort, toute création et toute suppression d'une juridiction de première instance. C'est une garantie de concertation avec les milieux judiciaires, les élus locaux- nous pourrions peut-être y rajouter les barreaux -, s'appuyant sur une évaluation publique, sans remettre en cause la compétence du pouvoir réglementaire. Pour faire face à ces inquiétudes, en particulier des fonctionnaires des greffes, nous avons prévu une garantie d'emploi au siège du nouveau tribunal ou au siège d'une chambre détachée, sous réserve d'une possibilité de délégation ponctuelle d'un fonctionnaire d'un site dans un autre, sur décision des chefs de juridiction. Cette garantie n'est pas nécessaire pour les magistrats, qui sont plus mobiles. D'ailleurs, il suffit de voir comment fonctionnent aujourd'hui les quelques chambres détachées qui existent en métropole. Nous nous sommes simplement fondés sur cette pratique.

La moitié des départements comportent plusieurs tribunaux de grande instance, et cette situation est un facteur important. Nous avons accepté certains de ces palliatifs : d'une part, la possibilité, et non l'obligation, pour le procureur général de désigner, vous l'avez rappelé, madame la ministre, un procureur chef de file, notamment pour les politiques partenariales, même si nous avons des doutes sur son application pratique, car cela exigera une coordination entre parquets ; d'autre part, la possibilité de ne pas avoir un juge d'instruction et un juge de l'application des peines dans chaque tribunal de grande instance. S'il est pertinent de renforcer le travail en équipe des juges d'instruction et de favoriser la cosaisine, la question semble moins évidente pour les juges de l'application des peines qui ont aussi une importante activité civile. Nous avons refusé un autre de ces palliatifs : la spécialisation, dans certaines matières civiles et pénales de grande technicité et de faible volumétrie, au sein d'un même département. La procédure nous paraît extrêmement lourde, pour des gains d'efficacité faible, dans des départements qui ne comportent que des petits tribunaux de grande instance, avec de faibles effectifs de magistrats, en supposant que les présidents de ces tribunaux parviennent à se mettre d'accord De plus, comment le justiciable pourrait-il s'y retrouver, alors qu'il ne sait pas à quel tribunal s'adresser ? En tous les cas, ce serait complexe. On risque, ce n'est pas exclu, de créer de nouveaux contentieux sur la compétence. Ces dispositions de spécialisation infradépartementale ne nous semblent pas utiles, sauf à vouloir- nous n'en faisons pas le procès -, à moyen terme, dévitaliser certains tribunaux sans le dire, mais dans ce cas, il aurait fallu aller directement au tribunal unique, ce sur quoi nous avions déjà débattu. Enfin, il reste la question du devenir du juge d'instance. Aujourd'hui, c'est une fonction spécialisée, c'est-à-dire que tout juge d'instance est nommé par décret dans un tribunal de grande instance pour assurer le service d'un tribunal d'instance donné. Même s'il peut participer à d'autres activités juridictionnelles, ce statut est une source de rigidité. Dans un premier temps, le Gouvernement a proposé de supprimer ce statut de juge d'instance, comme nous l'avions d'ailleurs suggéré nous-mêmes en 2017. Ainsi, seuls seraient spécialisées des fonctions relevant totalement ou en partie du champ pénal, compte tenu des garanties supplémentaires pouvant paraître nécessaires à cette matière, juge d'instruction, juge des libertés et de la détention, juge des enfants et juge de l'application des peines. Je rappelle que c'est d'ailleurs le Sénat qui, en 2001, a créé cette catégorie des fonctions spécialisées en les soumettant à des règles particulières de durée dans les fonctions. Pour assurer un traitement effectif et satisfaisant des contentieux de la vie courante, nous avions proposé, en 2017, de créer un juge chargé des contentieux de proximité. Nous avons repris cette proposition. Dans le cadre de l'ordonnance annuelle de roulement, le président du tribunal déléguerait des magistrats dans ces fonctions, tout comme pour le juge des affaires familiales. Ce magistrat pourrait alors siéger dans les chambres détachées et participer plus facilement aux activités du tribunal. en particulier aux audiences correctionnelles. Il semblerait que le Gouvernement a, quant à lui, changé d'idée. Il propose de maintenir le juge d'instance spécialisé sous le nom de « juge des contentieux de la proximité ». Outre que ce nom ne nous paraît pas complètement adapté au regard des compétences attribuées, une telle modification du projet de loi maintiendrait, dans l'organisation de première instance, une rigidité dans l'affectation des magistrats qui risquerait, au bout

Je partage, comme mon groupe, la position définie par la commission, mais je constate que les différences se sont réduites et je

: on observe toujours une grande différence entre ce que vous voulez faire et ce que les gens comprennent, entre ce que vous dites et ce que les gens entendent.

Marche, est ainsi libellé : La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à concrétiser une recommandation que notre collègue Richard Yung et notre ancien collègue Laurent Béteille avaient formulée, en 2011, dans leur rapport d'information sur l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon. Cette loi avait marqué une étape très importante dans la spécialisation des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle. Sur l'initiative de notre assemblée, elle avait notamment renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de confier une compétence exclusive en la matière à certains tribunaux. Le tribunal de compétent pour les brevets d'invention, les certificats d'utilité, les certificats complémentaires de protection et les topographies de produits semi-conducteurs. Par ailleurs, dix tribunaux de grande instance, dont celui de Paris, connaissent des actions relatives aux autres titres de propriété intellectuelle. Cette concentration de compétences présente de nombreux avantages : non seulement elle améliore le fonctionnement de l'institution judiciaire, mais elle est aussi un élément essentiel de rayonnement international du droit français et de l'attractivité juridique du territoire français dans un contexte de forte concurrence des systèmes juridiques nationaux. Il ressort de l'analyse du volume des dossiers traités par chacun des dix TGI spécialisés que cinq d'entre eux traitent moins de 5 % du contentieux de la propriété intellectuelle. Cette situation n'est pas satisfaisante au regard de la technicité du contentieux concerné et de l'impérieuse nécessité d'assurer une justice de qualité. Afin d'y remédier, nous proposons de réduire de moitié le nombre de TGI pouvant être désignés pour connaître des actions en matière de marques, de dessins et modèles, d'indications géographiques, d'obtentions végétales et de propriété littéraire et artistique. Ce renforcement de la spécialisation des juridictions civiles permettrait notamment d'harmoniser la jurisprudence. Pour ce qui concerne le contentieux marginal des obtentions végétales, il conviendrait de le confier au seul TGI de Paris

judiciaire indique que dix TGI sont toujours compétents pour connaître des actions en matière d'obtention végétale. Cela n'est pas raisonnable quand on sait que ce contentieux représente en moyenne une dizaine d'affaires par an.

fait le constat de l'insuffisance de la réponse pénale au phénomène de la contrefaçon ordinaire, c'est-à-dire des délits de contrefaçon autres que ceux qui présentent une grande complexité. Les juridictions répressives se voient toujours reprocher leur manque de fermeté tant sur les sanctions pénales que sur les indemnisations civiles. Cette timidité de la réponse pénale s'explique notamment par l'absence de spécialisation des juridictions répressives. Elle est par ailleurs la principale raison pour laquelle les juridictions répressives sont peu saisies d'atteintes aux droits de la propriété intellectuelle. Afin de remédier à cette situation préjudiciable aux titulaires de droits, nous proposons de confier à cinq tribunaux correctionnels une compétence exclusive pour le dossier simple de contrefaçon. En revanche, nous ne proposons pas de modifier le traitement pénal des affaires de contrefaçon présentant une grande complexité ; ces affaires continueraient de relever de la compétence des juridictions interrégionales spécialisées, conformément à l'article 704 du code de procédure pénale. Enfin, nous considérons que la mise en place de la disposition prévue dans le présent amendement devrait nécessairement s'accompagner de la création, au sein des juridictions spécialisées, d'une chambre mixte de propriété intellectuelle associant des magistrats civilistes et pénalistes. Une telle initiative permettrait selon nous une amélioration du dialogue des juges ainsi qu'une harmonisation des montants d'indemnisation versés aux titulaires de droits.

et que la quasi-totalité des requêtes en inscription est aujourd'hui déposée par voie électronique. Un établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé, l'EPELFI, a été créé à cette occasion. En lien avec les bureaux fonciers des tribunaux d'instance, l'EPELFI assure l'exploitation et la maintenance du système informatique qui a été conçu, ainsi que la sécurisation des données et de leur intégrité.

et du registre des associations coopératives de droit local. On permettra ainsi la consultation ou la réalisation des démarches à distance, à l'instar des dispositifs qui ont déjà été mis en place dans les autres départements pour les associations dites « loi 1901 ». Cet amendement vise à répondre à une demande de modernisation et de consolidation de l'informatisation de ces registres formulée par des acteurs locaux et relayée par le sénateur Jacques Bigot au travers d'un amendement n° 168. a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, mais la situation financière de l'EPELFI permettrait en réalité d'absorber cette nouvelle activité sans dépense nouvelle. En effet, la tenue des registres dont la gestion lui serait transférée est actuellement sous la responsabilité du ministère de la justice. Leur transfert à l'EPELFI, qui dispose déjà des fonds pour financer le projet et ne sollicitera donc pas de nouvelles contributions de la part du ministère de la justice, ne crée donc pas de charge nouvelle pour l'État, au contraire. Le Gouvernement a donc souhaité reprendre cet amendement à son compte, dans une rédaction plus aboutie. Les démarches des usagers seront ainsi facilitées, et les missions que les greffes des tribunaux d'instance d'Alsace-Moselle exercent au titre des registres des associations s'en

prolonger encore longtemps. En effet, vous le savez bien, tout droit qui n'évolue pas, qui ne se modernise pas, est condamné. Les Alsaciens-Mosellans souhaitent que leur droit local puisse continuer à être dynamique. Enfin, madame la garde des sceaux, je voudrais vous souhaiter plus de succès pour cet amendement que

cohérence dans les politiques conduites par les cours d'appel et de renforcer l'autorité judiciaire face à l'ensemble de ses partenaires régionaux. Peuvent être citées, à titre d'exemple, la mise en cohérence des procédures d'hospitalisation sous contrainte, en relation avec l'Agence régionale de santé, ou encore l'harmonisation des seuils de transactions douanières, avec la direction régionale des douanes. Cet article permet ensuite

Par rapport au projet initial du Gouvernement, l'amendement que je défends ajoute une précision importante : les matières qui pourraient donner lieu à cette spécialisation seront déterminées en tenant compte de leur technicité et de leur faible volume. Au fond, nous proposons au niveau des cours d'appel un mécanisme similaire à celui que j'ai exposé précédemment devant vous au niveau des tribunaux de grande instance. Ce dispositif fait donc qu'il n'est pas question d'expérimenter cette spécialisation pour des contentieux de masse. Cette expérimentation doit au contraire, en spécialisant les magistrats, permettre d'améliorer la qualité de la justice rendue dans les contentieux les plus techniques les plus techniques et donc de favoriser l'homogénéisation de la jurisprudence au niveau régional. Les conclusions de cette expérimentation seront transparentes ; un rapport complet sera remis au Parlement. Je vous demande donc de bien vouloir rétablir l'article 54 dans la version que vous propose ici le Gouvernement.

une utilité réelle semble-t-il, à développer une forme de hiérarchisation implicite entre les cours, qui existe déjà en matière budgétaire et qui n'est pas réellement acceptée, à supposer que les chefs de cour s'y prêtent. En matière budgétaire, il existe aujourd'hui, dans le cadre du dialogue de gestion avec la direction des services judiciaires, des cours responsables du budget opérationnel de programme- connu sous le sigle BOP -et d'autres, simples unités opérationnelles. Mais cette distinction ne se traduit pas par une réelle hiérarchisation, laquelle ne serait pas tout à fait acceptable, les cours disposant pour l'essentiel des mêmes compétences juridictionnelles.

ils font un travail formidable, tout en étant trois fois moins payés que des avocats. Pour autant, le risque de contestation de ce système est latent. Il n'y a aucune raison pour que les habitants de Wallis-et-Futuna n'aient pas droit à des avocats commis d'office, comme les citoyens de métropole, dans le cadre de l'aide juridictionnelle Je suis bien conscient qu'aucun avocat ne souhaite ouvrir un bureau à Wallis, et que les avocats du barreau de Nouméa ne se bousculeront pas pour faire plusieurs heures d'avion et, surtout, rester bloqué deux ou trois jours à Wallis, puisque nous ne sommes desservis que par deux vols par semaine. Reste qu'il est aujourd'hui

J'espère, madame la garde des sceaux, qu'il vous sera possible de tenir compte de cette remarque importante dans le cadre des ordonnances que votre ministère va préparer, afin de faire progresser la question de l'aide juridictionnelle à Wallis-et-Futuna. Je suis saisie

Nous sommes évidemment opposés à cet article, pour diverses raisons. La première est le recours à la procédure de l'article 38, qui dessaisira le Parlement de son rôle dans la confection de la loi au profit d'une concertation limitée, dont les participants ne sont pas connus et dont les motivations sont éloignées de l'intérêt général. Notre opposition sur la forme à la procédure de l'article 38 résulte également de la tendance importante observée ces trois derniers quinquennats à un recours aux ordonnances de plus en plus élargi. Comme si la procédure d'habilitation était devenue, avec la procédure accélérée d'examen des projets de loi, l'une des armes fatales de l'exécutif face au possible renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement à la suite de l'application concrète de la session unique. Ce sont ainsi plus de 500 projets de loi potentiels qui ont été transformés en ordonnances au cours de chacun des deux derniers quinquennats. L'actuel prend le même chemin. En ce qui concerne la modification à venir de la carte judiciaire, les craintes les plus sérieuses peuvent naître de la technocratie en action, transformant la présence territoriale de nos tribunaux en algorithmes plus ou moins obscurs, qui ne valideront par avance qu'une présence obligée des services judiciaires et juridiques. la carte judiciaire participe de l'aménagement du territoire. Toutes les évolutions qu'elle pourrait subir conduisent naturellement à s'interroger sur le sens que l'on peut donner à cette notion d'aménagement du territoire, comme au respect de l'un des principes républicains les plus essentiels : l'égalité d'accès aux droits, contrepartie naturelle de la participation des citoyens au financement de l'action publique. Mettre en cause la carte judiciaire,

pour tirer les conséquences de la création de ce nouveau juge spécialisé. Cet amendement a en outre pour objet de restaurer la référence au tribunal de grande instance, le maintien de cette dénomination permettant, ainsi que je l'ai déjà expliqué, de conforter la lisibilité de notre organisation judiciaire.

d'un amendement quasi rédactionnel. Il vise en effet à supprimer la précision selon laquelle les modifications apportées par l'article 55 à l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution auraient un caractère interprétatif.

en charge de la construction de la prison et de l'intégration des gardes dans l'administration pénitentiaire par le biais du dispositif de la loi Sauvadet. Vos réponses, madame la garde

Bien que la justice soit une compétence régalienne, la gestion du service pénitentiaire à Wallis-et-Futuna fait l'objet d'une convention de 1997 entre l'État et le territoire. Le principe en est que le territoire avance les frais de fonctionnement et que l'État les lui rembourse.

mission envisageait la prise en compte du service pénitentiaire par le ministère de la justice pour le 1 janvier 2019. madame la garde des sceaux, et surtout des fonds engagés sur le budget territorial qui n'ont pas encore été remboursés ? La créance du territoire entre 2011 et fin 2017 s'élève à plus de 19 millions de francs, soit environ 160 000 euros, une somme importante pour un petit territoire comme le nôtre. Madame la garde des sceaux, la justice demeure une mission régalienne par excellence : elle ne saurait incomber aux collectivités territoriales

Les délais de mise en oeuvre du programme immobilier pénitentiaire nécessitent de reporter le moratoire sur l'encellulement individuel à 2022 sur le territoire de la République dans son ensemble, y compris les îles de Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Une disposition expresse doit